La parole est à monsieur Antoine Lefèvre pour une mise au point, au sujet d'un vote. Oui, merci monsieur le président, mes chers collègues, je souhaite faire la mise au point suivante sur le scrutin public numéro 119. Mon collègue Philippe Paul et moi-même souhaitons nous abstenir merci. Merci cher collègue. Donner de cette mise au point sera publié au Journal officiel et figurera dans la liste politique du scrutin monsieur Jean-Michel Arnaud veut aussi faire une mise au point sujet dans votre. Je vous remercie. Je souhaite effectivement fait hein de réification de vote concernant. Olivier Cadic. Concernant le scrutin numéro 119 séance du 1er février 2023. Pourtant, sur l'amendement numéro un rectificatif bis présenté par Philippe Bas. Monsieur Olivier Cadic a indiqué vouloir voter pour donc rectification de vote donné, merci. J'informe le Sénat que les candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie de la santé, du travail des transports et de l'agriculture ont été publiés. C'est quand dictature seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à renforcer l'action des collectivités territoriales en matière de politique du logement présenté par Monsieur Ronan Dantec et plusieurs de ses collègues. Demande du groupe écologiste solidarité et territoires. La discussion générale. La parole est à monsieur Ronan Dantec, auteur de la proposition de loi pour 10 minutes.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur. Monsieur le président de commission. Je voudrais tout d'abord partager avec vous ma conviction profonde. Les difficultés d'accès au logement sont aujourd'hui un des principaux facteurs peut être le principal de la déstabilisation de la société française, cette conviction et celle des sénatrices et sénateurs du groupe écologiste qui ont tenu à mettre une PPL une proposition de loi sur le logement dans leur niche mais elle est je crois partagé sur tous les bancs par des sénateurs de différentes régions tous confrontés à l'accélération de cette fracture ce sentiment d'injustice ses difficultés au quotidien pour se loger nourrissent l'aigreur collective le vote pour une offre extrémistes de recroquevillée. Néanmois et c'est la bonne nouvelle du moment, toute la France ne se résigne pas aux injustices sociales. Les manifestations de ce mardi l'ont montré. Le coût du logement n'a cessé d'augmenter de manière considérable depuis 30 ans. Le phénomène et s'installe d'abord dans les zones urbaines à Paris et en petite couronne dans les années 90, puis dans les métropoles comme par exemple Nantes RN dans les années 2000 ou Bordeaux. 10 ans plus tard, il n'est pas si rare de voir aujourd'hui des bien se vendre en euros au même prix qu'il y a 30 ans. Mais à l'époque, c'était en franc, une multiplication par six en 30 ans. Nous connaissons les conséquences de ce déséquilibre en terme de reflux de la mixité résidentielle et scolaire Éric Maurin, on parlait déjà il y a 15 ans d'étalement urbain d'explosion des mobilités contraintes et de la consommation d'espaces naturels et agricoles. La nécessité et l'urgence Dusan du zéro artificialisation nette est ainsi en lien Direct avec cette ruptures dans les parcours résidentiels pour les petites classes moyennes et leur éloignement des centres urbains. Ces 30 dernières années et la crise du Covid là semble-t-il encore accélérer la ruée vers les zones littorales de l'Ouest et du Sud-Ouest et l'augmentation vertigineuse des prix de l'immobilier en bord de mer. Oh aussi entraîné une véritable fracture dans le peuplement. Je suis d'origine finistérienne, nous ne pouvions pas imaginer que dans ce département où les habitants sont particulièrement attachés à leur commune. Il deviendrait en 5 ans à peine, impossible pour beaucoup d'acquérir une maison même petite sur leur territoire de naissance et de vie et le sénateur de Atlantique que je suis ne peut que constater la situation inextricable dans un département qui cumule attractivité métropolitaine et attractivité touristique dans ce département, c'est maintenant vers les départements limitrophes que sont pousser les ménages modestes avec les difficultés que nous savons en termes de mobilité et d'accès aux services publics et je ne parle pas ici de tout ce qui ne trouvent tout simplement plus à se loger. Les chiffres publiés par la Fondation Abbé Pierre sont suffisamment éloquents à ce sujet et je souligne que la fondation insiste notamment sur l'explosion du mal logement en zone littorale. Nous sommes donc dans une situation grave et le débat des jalons que nous avions eu lors du projet de loi de finances. Monsieur le président, avec des cris d'alerte venant de tous les bancs de cet hémicycle, a souligné l'urgence à agir. Cette proposition de loi n'a pas la prétention de régler à elle seule la crise actuelle courte c'est quand même une PPL elle veut d'abord souligner l'importance de l'intervention des collectivités territoriales sans lesquelles nous ne pourrons agir efficacement. Elle propose donc d'en renforcer les Budgets pour conforter l'action les régions tout d'abord. Elles ont acquis depuis la loi notre une compétence pour fac-similés l'accès au logement. Certaines sont sont d'ailleurs saisi pour financer, même la production de logements sociaux. Mais c'est surtout le sera d'être le document de planification régionale dont elles ont la charge qui va devenir de plus en plus le document stratégique de référence qui fixera les lieux de la production de logements car il intégrera notamment monsieur. Le rapporteur. La cartographie de synthèse Dusan après les travaux menés à l'échelle des plus pays à lui La région va jouer un rôle de plus en plus important dans les politiques de logement indissociable des politiques d'emploi et d'aménagement du territoire. C'est le sens de l'histoire, elle se doit donc d'être conforté, car ce besoin en ingénierie en animation territoriale, sans parler des aides directes à la construction vont être de plus en plus important. Je n'ignore pas qu'il y a au sein des régions. Une difficulté aujourd'hui dans la manière de décliner cette compétence sur l'accès au logement, nous le savons. Certaines régions sont réticentes à se positionner plus fortement sur cette compétence au risque d'être happé et de se retrouver demain en première ligne. cette modeste PPL participe du débat nécessaire sur ce rôle des régions dans les futures politique du logement et d'après certains échos sur les débats qui a sollicité cette PPL il n'était probablement pas inutile de mettre déjà une pièce dans la machine. Beaucoup plus consensuel, le renforcement du rôle des établissements publics fonciers locaux les EPFL est souhaitée par tous. Je ne connais pas aujourd'hui en Loire-Atlantique. Un seul élu, quelle que soit sa couleur politique qui ne le demande pas et vous avez d'ailleurs reçu chers collègues un courrier de soutien très clair du réseau des EPFL à cette proposition de l'eau. Je ne suis pas rentrer dans cette PPL sur l'articulation entre EPFL et EPF eux entre les établissements publics fonciers locaux gérés directement par les intercommunalités et les États maison public foncier d'État où il y a quand même bien sûr aussi un rôle important des collectivités locales. Le débat, il était trop large mais il devra être tenu. Nous avons simplement cherché avec mes collègues du groupe écologiste à répondre à l'urgence, sachant qu'avec la mise en oeuvre Dusan les besoins d'intervention sur la réhabilitation des corps goût ou sur d'anciennes zones artisanales. Économiques vont devenir de plus en plus considérable d'ores et déjà, je prends l'exemple de la Loire-Atlantique malgré son renforcement. L'EPFL ne peut pas déjà répondre à l'ensemble des demandes des communes. Cette propositions cet article de de notre proposition de loi devrait donc, je crois, faire l'objet d'un véritable consensus entre nous et nous permettent de gagner du temps parce que si on la vote il y a évidemment après évidemment encore la navette parlementaire. Ça veut dire déjà que le temps que les EPFL vote des changements de taux si elle le souhaite, ce que je rappelle que cette proposition passe par l'optionnel, enfin ça va mais déjà un an ou 2 ans, donc on voit bien que par rapport à l'urgence. Il s'agit maintenant véritablement de gagner du temps. Mais qui dit dépenses. Pour les régions ou pour les EPF elle dit recettes. À l'inverse, c'est toujours le la partie du débat qui est à moins consensuel. La logique de cette PPL et donc d'asseoir les recettes sur un des facteurs de déstabilisation actuel qui est l'explosion du nombre de résidences secondaires dans certains territoires. Aujourd'hui, le nombre de résidences secondaires, augmentent plus rapidement que la production de logements neufs c'est prêt par exemple de 300.000 résidences secondaires en Bretagne aujourd'hui. C'est donc un facteur de déstabilisation et je regarde mon collègue Max Brisson. La situation du Pays basque. On est totalement caractéristiques. il est clair que les résidences secondaires participe de la déstabilisation du marché du logement en ajoutant donc une soeur raisonnable de 0 à 25% pour les propriétaires de ces biens. Nous ne les amèneront probablement pas les remettre sur le marché. C'est pas le sens de cette PPL mais nous permettront une augmentation substantielle de la capacité d'action des EPFL qui pourraient dans certains territoires en appliquant le 25% voir leurs recettes. D'après nos calculs, multiplié par 2, nous avons limité aux zones tendues puisque c'est les zones où les résidences secondaires joue un rôle de déstabilisation. Le plus important mais je pense qu'effectivement le débat est ouvert pour aller sur la totalité des périmètres des EPF Enfin, et j'insiste beaucoup sur ce point, il s'agit d'une possibilité non d'une obligation, ce sont les élus qui gèrent les EPFL qui décideront, ou pas, de cette augmentation augmentation que nous avons donc voulu extrêmement raisonnables, entre 0 et 25%. Nous avons repris une proposition votée ici au Sénat, porté à l'époque, c'était il y a quelques semaines par Philippe Bas. Je ne sais pas s'il faut prendre Philippe Bas en exemple. Ce matin, mais en tout cas cette proposition avait fait quasi-consensus. Dans l'hémicycle. Donc, nous, une somme en fait. Inspiré de ce que vous avez déjà voté, chers collègues. Le Sénat regrette très régulièrement la perte d'autonomie fiscale des collectivités. C'est un autre point de consensus entre nous. Cette proposition de loi la renforce tout simplement. Le Sénat s'émeut de la déstabilisation du marché du logement en zone littorale avec de nombreuses interventions dans cet hémicycle. Cette proposition de loi propose de renforcer l'action des élus locaux pour y répondre n'ayant une proposition de loi qui s'est beaucoup inspiré des débats les plus consensuel que nous avons eu dans cet hémicycle, nous ne pouvons qu'espérer un vote largement majoritaire sur une proposition simple, qui s'inscrit d'abord dans l'urgence. Je vous remercie. Merci cher collègue. Là. Parole est à monsieur Jean Baptiste Blanc, rapporteur de la commission des finances pour 10 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre et mes chers collègues, nous avons assez longuement débattu dans le cas du dernier projet de loi de finances au sujet du développement des résidences secondaires. Et de ses effets sur le marché local de l'immobilier en particulier sur les contraintes en termes d'accès au logement pour les résidents permanents. Depuis 2010, on constate une accélération assez nette du nombre des résidences secondaires qui a augmenté de 16 et demi pour 100, contre moins de 10% pour les résidences principales. La proportion de résidences secondaires est particulièrement élevée sur le littoral Atlantique en effet et en Corse. Ce développement accentue la tension sur le marché du logement et surtout dans les territoires où la population est en augmentation, obligeant les personnes travaillant dans les communes touristiques a résidé elle-même de plus en plus loin. Il faut toutefois se garder d'une vision uniforme selon laquelle le développement des résidences secondaires seraient systématiquement défavorables aux résidents locaux. Les résidences secondaires constituent aussi une source d'attractivité et d'enrichissement pour l'économie locale en particulier là où la densité de population est moins importante face à ce phénomène et la fiscalité locale a évolué significativement ces dernières années en faveur des résidences secondaires par rapport aux résidences principales, je rappellerai de mesures. La première, la taxe d'habitation a été supprimée progressivement sur les résidences principales. Depuis le 1er janvier 2023 ne s'applique qu'aux seuls résidents secondaires. D'où son appellation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires Th RS. En second lieu, la loi de finances pour 2023 a étendu le périmètre dans lequel s'applique à la fois la taxe sur les logements vacants et où les communes peuvent également appliquer une majoration de 5 à 60% de la taxe d'habitation des résidences secondaires. Ce périmètre se limitait auparavant à des zones tendues de plus de 50.000 habitants. Est désormais la majoration de TH RS pour être décidée dans des communes situées dans des zones d'urbanisation plus petites, notamment celles où le taux de résidences secondaires est élevé. La liste de ces communes et ce n'est certes pas encore connu. Car le décret d'application, Monsieur le Ministre, n'a pas été pris. Peut-être serez-vous en mesure de nous apporter aujourd'hui des précisions sur un éventuel calendrier relatif à ce décret. Lorsque le nouveau zonage sera connu des milliers de communes acquerront probablement la possibilité de majorer la tâche R. T hrs précisément dans les zones visées par la présente, proposition de loi. Le développement des réseaux secondaires et donc un phénomène avéré qui doit être prise en compte dans les politiques du logement. La proposition de loi que nous examinons et des des déposée par Monsieur Ronan Dantec, et les membres du groupe écologiste solidarité et territoires Ronan Dantec. Que je salue la qualité de son travail. Je salue la qualité de nos échanges, j'associerai Daniel Breuiller anneaux ce compliment. J'ai Ronan donc en tout cas la PPL constate ce phénomène et cherche à apporter à certaines catégories d'acteurs publics, à savoir les régions, les établissements publics fonciers locaux les moyens d'accomplir leur mission en matière de politique du logement et l'aménagement. Les 2 Arctique sont similaires dans leur dispositif il s'agit de créer de taxe additionnelle à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. La première serait instituée au profit de la région sur délibération du conseil régional, c'est donc l'article 1er, la seconde serait reversée aux établissements publics fonciers EPF locaux et à l'Office foncier de Corse, c'est l'article deux. Dans les deux cas, ce n'est pas l'ensemble du territoire qui est visée mais les zones dans lesquelles. Peut s'appliquer la taxe sur les logements vacants et la surtaxe CHRS, c'est-à-dire les zones tendues, notamment touristiques en outre la taxe l'article de ne s'appliquerait que dans le périmètre des EPF locaux. C'est-à-dire sur une part très limitée du territoire national, car la plupart des territoires sont couverts uniquement par un EPF d'État voir aucun EPF il y a des zones blanches, nous le savons tous les fraudeurs. D'ailleurs, traiter ce problème. Le taux de chacune de ces taxes pourraient varier de 0 à 25% de la valeur locative en fonction des délibérations du conseil régional ou du conseil d'administration de l'EPF comme l'indique l'exposé des motifs, il s'agit d'abord de taxe de rendement qui vise à apporter des ressources aux régions et aux EPF locaux. Aurait-elle une influence sur les les propriétaires de résidence secondaire, cela est difficile à déterminer. On peut penser que beaucoup d'entre eux ne vont pas mettre en location de manière permanente, un logement simplement parce que le taux de taxation aura augmenté, il est possible toutefois que certains fassent le choix d'acquérir une résidence secondaire dans une zone où ces taxes ne seront pas instituer ce qui pourrait donc avoir un effet sur la politique de logement local. Or l'un des principaux obstacles que je vois ces dispositions est celui de la mise est celui de la mise en cohérence entre les autorités en charge de la compétence. Logement et d'un côté, si l'État conserve une part essentielle dans la définition de la politique du logement, notamment dans les aides de guichet, la mise en oeuvre locale de la politique du logement relève pour l'essentiel des communes et des intercommunalités. Même si la loi notre a attribué aux régions une compétence pour promouvoir je cite le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine. S'agissant des EPF. Cette proposition de loi leur permettrait non seulement d'accroître leurs ressources mais aussi, et ceci est une nouveauté de décider sur quelle catégorie de contribuables cette ressource serait prélevée en l'occurrence et les propriétaires de résidences secondaires. Je crains donc qu'il y ait un risque d'interférence ou de manque de cohérence dans la mise en oeuvre de la politique de logement car les régions et les EPF d'une part et les communes et intercommunalités, d'autre part non, ni le même périmètre, ni nécessairement les mêmes stratégies de surcroît cette ressource était assortie d'aucune obligation d'utilisation et rien ne garantit donc que le leur, leur produit dans le cas des régions seraient effectivement utilisé pour les actions en faveur de l'accès au logement. D'ailleurs, les régions ne sont pas demandeuses de cette ressource du point de vue du contribuable. Les nouvelles taxes et la hausse brutale de la taxe d'habitation qu'elles entraîneraient serait importante. Logement taxé aujourd'hui à 30 ou 40% pourraient être taxés désormais à 80 ou 90% avec l'ajout de nouvelles lignes sur l'avis d'imposition qui rendrait plus difficile encore la compréhension de la fiscalité par les contribuables. Le risque d'inconstitutionnalité liés à de tels taux d'imposition et d'ailleurs, élevé en application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. En outre, comment justifier du point de vue du principe d'égalité entre les contribuables que la taxe prévue par l'article de puisse frapper le logement situé dans le périmètre. D'un EPF local mais pas celui qui est située dans le périmètre d'un EPF d'État pour l'ensemble de ces raisons, la commission des finances n'a pas adopté cette proposition de loi et vous proposera donc le rejet de ces 2 articles la solution paraît en effet prématuré voire d'adapter même si le sujet soulevé est réelle, je le redis. Par exemple il paraît nécessaire de permettre aux établissements publics fonciers d'assurer leur mission qui iront croissant au cours des années à venir les EPF participe au programme Action coeur de ville Petites Villes de demain à la réhabilitation à la dépollution de friches à la constitution de réserves foncières pour les collectivités. De manière générale, la mise en oeuvre du zéro artificialisation nette va entraîner mécaniquement une raréfaction de la ressource foncière. Il est important que les collectivités puissent s'appuyer sur les EPF or les EPF sont en partie financé par une dotation budgétaire qui compense en effet. Qui compense pardon les effets de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, faut-il maintenir cette dotation qui ne prend pas en compte les extensions de périmètres des EPF la renforcer ou au contraire envisager de ressources fondée sur une assiette locale et moins soumise aux arbitrages annuelle de l'État. Voilà l'une des questions sous-jacentes à cette proposition de loi, la réponse n'est probablement pas dans la création de nouvelles taxes surtout réservé à une catégorie de PF la taxation des raisons secondaire doit s'apprécier dans un périmètre plus large, qui est celui du financement de la politique locale du logement et de l'aménagement. Et par ailleurs, si nous devons laisser vivre les évolutions de la fiscalité proposée par la loi de finances pour 2023, c'est-à-dire la possibilité de majorer la tâche. Hrs qui va être précisément aux territoires visés par cette PPL en outre les conditions concrètes de la d'application du doivent évoluer avec la révision des décrets pris l'an l'an passé et nous l'espérons, une évolution du cadre légal, telle que la propose. La proposition de loi visant à faciliter la mise en oeuvre objectif Dusan au coeur des territoires pour laquelle le Sénat vient de constituer une commission spéciale hier. il faudra en s'appuyant sur des travaux tels que le récent rapport du Conseil des prélèvements obligatoires sur la fiscalité Dusan. Avancer sur la définition de la fiscalité et du financement de cet objectif. Je vous remercie. La parole est à monsieur Franck re-Riester Ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le président. Monsieur le président de la commission des finances. Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs. Le texte examiné ce matin permet de mettre en lumière un phénomène particulièrement prégnant dans de très nombreux points de notre territoire. Le constat que vous établissez monsieur le sénateur Dantec est en effet d'une très grande clarté et d'une très grande justesse. L'inflation des prix de l'immobilier alimenté notamment par la multiplication des résidences secondaires. Crée un problème d'accès au logement pour les Français qui parfois depuis des générations. Vivent dans ces villes dans ces départements dans tous les lieux touchés par ce phénomène est particulièrement bien sûr dans la région qui est la vôtre, monsieur sénateur. Les chiffres de l'Insee en atteste cette tendance s'est accélérée au cours de la dernière décennie. Depuis 2010 le nombre de résidences secondaires a augmenté de 16,5%, contre moins de 10% pour les résidences principales. Même si les résidences secondaires représentent environ un logement sur 10. Il faut être attentif à la dynamique à l'heure. Et cette multiplication des résidences secondaires ne concerne pas uniquement le sud de la France mais aussi la côte Atlantique et les agglomérations de grandes métropoles comme Lyon, Toulouse ou encore Bordeaux. Le gouvernement partage donc une très grande partie du diagnostic que vous dressez. Les tensions sur les prix sont incontestables et certaines communes ou quartiers sont devenus inaccessibles pour des gens qui doivent alors déménager pour aller vivre plus loin. Plus loin de leur travail plus loin des lieux dans lesquels ils sont parfois n'est plus loin des lieux auxquelles ils sont profondément attachés. Et ce d'autant que ces zones souvent touristique se dévitaliser en ne connaissant plus que des habitants intermittents à mesure que les résidences secondaires deviennent prépondérantes. Votre PPL pose ainsi des questions sérieuses de très nombreux parlementaires sénateurs mais aussi députés ou élus locaux se retrouvent sans doute dans le constat que vous faites. Pour y répondre vous proposer des mesures de nature fiscale. Sans conteste la fiscalité plus largement l'incitation financière. A son rôle à jouer mais elle doit d'être. En complément d'autres instruments et ne peut à elle seule tout résoudre. De façon générale, le gouvernement a la conviction qu'on ne peut pas régler tous les problèmes de notre pays par une accumulation de taxes ou d'impôts et qu'en cette période, nous devons collectivement veiller à ne pas multiplier les prélèvements sur nos compatriotes. D'autant que les résidences secondaires ne sont pas forcément détenues par les plus aisés. Insee estime que 34% des propriétaires de résidences secondaires appartiennent au dernier décile de la distribution de revenus. Car, concrètement c'est PPL propose de créer de nouvelles taxe additionnelle à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Dont les recettes bénéficieraient respectivement aux régions et aux établissements publics fonciers d'État et locaux. Cette taxe s'appliquerait dans les zones géographiques en tension qui conditionne déjà la possibilité pour les communes d'appliquer une majorité majoration de la TH RS. La première tac serait institué sur délibération du conseil régional qui pouvaient en fixer le taux dans une fourchette comme vous l'avez évoqué, monsieur le sénateur comprise entre 0 et 25% de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires qui s'applique dans la commune concernée. La seconde obéit à un mécanisme similaire mais celle-ci serait instituée au profit des établissements publics fonciers. Alors le gouvernement ne peut soutenir cette proposition pour plusieurs raisons. D'abord, et je l'ai évoqué tout à l'heure parce que le gouvernement est très attentif à maîtriser la pression fiscale dans notre pays. On vous proposer un cumul d'imposition qui pourrait d'ailleurs être considéré comme confiscatoire par le juge constitutionnel. En effet, une même assiette fiscale en l'occurrence la valeur locative cadastrale d'un bien. Se verraient appliquer une succession de taxes et de majorer et de majoration avec au final un taux d'imposition globale à des niveaux extrêmement élevés. À titre d'illustration, le taux d'imposition pour les résidences secondaires situées à Grenoble pourrait atteindre plus de 84%. Nous doutons que le Conseil constitutionnel puisse valider cela. J'ajoute que le type de fiscalité que vous proposez existe déjà largement puisque les établissements publics fonciers par exemple. Perçoivent déjà des taxe spéciale d'équipement répartis sur les impôts fonciers dont la TH RS. justement des établissements publics fonciers locaux la TSE est fixé par les établissements en fonction de leur engagement financier dans la limite de 20 euros par habitant. En pratique, il demeure une marge significative. Sous ce plafond car le montant moyen de la TSE et tu. De 11 euros sur l'ensemble du territoire aujourd'hui. En termes de financement des établissements fonciers. Nous estimons donc que des marges existent sans créer de nouveaux prélèvements. Deuxièmement, parce que l'outil que vous recherchez existe déjà et que nous avons beaucoup avancé sur ces sujets dans le cadre de la dernière loi de finances. Tout d'abord je veux rappeler qu'en 2023 et le gouvernement s'en félicite. La taxe d'habitation est intégralement supprimée sur la résidence principale mais continue de s'appliquer sans aucune autre forme d'allégement pour les résidences secondaires. Cette réforme crée donc un différentiel de fiscalité qui permet de rendre fiscalement bien plus attractive, l'occupation d'un logement en tant que résidence principale. Surtout dans le cadre de la loi de finances pour 2023, nous avons renforcé les marges de manoeuvres dont disposent les communes pour imposer les résidences secondaires. À l'initiative du député, Xavier Roseren. Dont la proposition a été approuvée par le Sénat, la définition des zones tendues, a été complété pour intégrer pleinement les communes touristiques dans le Champ de cet outil en cas de tension. C'est un levier extrêmement puissants dans les zones en tension le les logements vacants sont automatiquement imposer la taxe sur les logements vacants. Après un an de vacances ou les conseils municipaux peuvent décider d'instituer une majoration de la cotisation de ta TH RS comprise entre 5 et 60%. J'ajoute que toujours dans cette optique de résorption de la non occupation des logements. La dernière loi de finances a augmenté d'un tiers les taux de la télé. à compter 2023 les taux de la TV sont portés à 17% la première année et 34% dès la 2ème au lieu de 12 ennemi et de 25 jusqu'à pour Ce sont des outils extrêmement puissants, je le disais à titre d'exemple, appliquer la majoration hauteur de 60%, représentent un montant d'impôt de 536 euros pour. Par un appart

Cette réforme assure que des communes qui présente une part de résidences secondaires très significative pourront activer ce levier alors que ce n'était pas le cas aujourd'hui. Lorsqu'elle ne faisait pas parti d'une aire urbaine ou que le niveau de tension sur le marché locatif était un peu moindre que dans les zones les plus tendues du territoire. En cela je crois que la réforme répond directement aux aspirations d'un grand nombre d'élus et de territoire, notamment dans les halles en Corse sur le littoral Atlantique et méditerranéen. Et en Bretagne. C'est aussi une réforme qui conserve le principe d'un zonage territorial pour éviter une augmentation fiscale indiscriminées. Le gouvernement travaille en ce moment même en concertation avec les associations d'élus. À l'élaboration du décret d'application de cette réforme qui précisera les zones d'application. Vous l'avez évoqué, monsieur le rapporteur. Tout à l'heure. Je sais que certains d'entre vous ont pu être interpellés sur le fait que les communes ne pourront pas dès cette année percevoir la recette liée à l'application de cette Marache majoration. Je tiens à vous rassurer sur le fait que ce décret sera pris dans les meilleurs délais délai et permettra aux communes entrantes, avant le premier octobre prochain de délibéré pour majorer la TH RS à compter des impositions de 2024. Aussi, Monsieur le Sénateur. Les objectifs de cette réforme introduite en loi de finances pour 2023 sont très largement convergentes avec le texte que vous proposez. Elle renchérit l'occupation de résidences secondaires dans les zones qui sont saturés et ce dans des proportions très significative. Elle permet de procurer de nouvelles ressources communes pour exercer leurs compétences en matière d'aménagement du territoire. Assurer une offre de service public malgré la déprise des résidents permanents et financer des projets immobiliers qui concourront au rééquilibrage que vous appelez de vos voeux. Ces communes pourront aussi faire le choix d'utiliser ce produit supplémentaire. Pour augmenter leur contribution aux établissements publics fonciers. Vous le voyez, c'est une réforme qui répond de façon ciblée et proportionnée aux enjeux de la rétention foncière l'accès au logement. En rappelant ses éléments je ne veut toutefois pas laisser penser que le gouvernement fait de la fiscalité l'Alpha et l'oméga pour orienter le marché immobilier. Une partie du phénomène d'attrition de logement que vous décrivez est lié au rôle des plateformes de locations de courte durée qui ont permis de démocratiser cette activité au détriment de l'offre hôtelière. Les études disponibles montrent un impact à la hausse des prix de l'immobilier au fur et à mesure de la croissance de l'activité de location de courte durée et une diminution des locations longue durée par substitution. On constate aussi que ces locations brèves tendent à devenir plus intensive donc à se professionnaliser et qu'elle se concentre sur des biens qui constitue la première étape d'un parcours résidentiel en habitation principale pour les plus modestes, à savoir les biens de moins de 40 m2. Depuis Depuis la loi Elan nous avons institué un cadre réglementaire ambitieux pour essayer de maîtriser ce phénomène. Cela passe en particulier par la réglementation du changement d'usage qui ouvre ensuite un droit de compensation pour les communes ne se sont toutefois pas encore suffisamment saisi. C'est tout le sens de la réflexion que mène en ce moment même. Dominique Faure et Olivia Grégoire sur ce sujet. Je ne serai pas plus long sur ces questions qui vont au-delà de votre proposition de loi, mais qui montre que le gouvernement s'est saisi du sujet que nous devons avoir sur ces questions essentielles, une approche qui ne se cantonne pas la fiscalité mais je sais que c'est aussi votre volonté. Vous l'avez compris, pour toutes ces raisons, l'avis du Gouvernement sera défavorable sur cette proposition de loi en raison des moyens que vous proposez pour atteindre un objectif auquel, en revanche le gouvernement souscrit pleinement. Je vous remercie. Si Monsieur le Ministre, dans la discussion générale. La parole est un président Jean-Claude Requier pour le groupe RDSE pour 4 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la caution finances monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. L'intention de cette proposition de loi de notre collègue Ronan Dantec. Et tout à fait louable. L'accès au logement et en particulier la possibilité de demeurer dans son lieu de naissance de vie et l'attachement. Sont des enjeux majeurs encore aujourd'hui en France en 2000 Les questions de logement, quel que soit le point de vue qu'on adopte son petit éminemment sensible. On le voit cette semaine avec l'examen concomitante de cet hémicycle de la proposition de loi sur l'occupation illicite mais aussi de la situation de certains locataires. Tout à fait licite.

C'est un fait connu que la fouille des populations à fort pouvoir d'achat un territoire donné tant à chasser les premiers occupants ou leurs descendants souvent incapables de fuir financière. L'attachement à ce territoire de naissance ou de jeunesse. Reste fort dans notre beau pays malgré les bouleversements de la vie moderne. Je dirais même plus, la perte de repères est forte, plus paradoxalement le besoin d'enracinement et grand. J'ajouterai que le phénomène ne se limite pas aux zones côtières dans le Sud-Ouest on était si habitué à la présence ancienne. De résidents d'origine britannique. Soit à fort pouvoir d'achat. Même si le Brexit a rendu leur situation plus compliquée. Les auteurs de la PPL dit vouloir préserver. Le droit de vivre dans le territoire de l'essence et de lui. Face à un marché du logement est suffisamment réduit. Nul doute que le marché immobilier souffrent de défaillances. En témoignent les difficultés de mise à l'heure de l'encadrement des loyers dans les zones tendues. Par ailleurs, la spéculation immobilière et foncière est une réalité qui pèse lourdement sur beaucoup de nos concitoyens. Inversement, dans les territoires en perte fluide d'attractivité la Rowan bien à prix raisonnables peut être difficile pour autant la réponse apportée par la PP avait été adéquate. On peut en douter. Dans la mesure où elle entend répondre à ces enjeux par la création de de taxes. D'abord le rétablissement une taxe régionale sur les résidences secondaires, elles auraient pour objectif de renforcer la capacité d'animation territoriale des rayons. En matière de logement. Il y a des compétences et des dispositifs existants comme le développement économique et les schémas régionaux d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires et le fameux Stradella. Ensuite une taxe additionnelle à la taxe a lieu d'habitation ni rien secondaire la TH RS. Au profit des des gens foncier d'État et locaux qui leur permettrait de préempter des biens immobiliers dans une optique de rééquilibrage territorial. À l'instar du rapporteur, j'ai mes DVD annonce la création d'un boulot, la pression fiscale manière générale étant donné la forte. Par ailleurs, on observe déjà l'augmentation des taxes foncières. Depuis la suppression de la TH sur les Real ce principal a su qui peut nous assurer que ces ressources. Source servirait réellement à financer les politiques indiqué alors que la taxe d'habitation ne subsiste plus que sur les réseaux secondaires. On a vu la dernière finale les difficultés engendrées. Pour les collectivités

Monsieur le président, Monsieur le Ministre. Monsieur le monsieur le président. La commission des finances, monsieur le rapporteur. Chers collègues. Les constats sur les difficultés des ménages à se loger sont connus. Ce problème public fait régulièrement la une de l'actualité et des travaux parlementaires. Lors de, d'un débat sur la crise du logement à l'initiative de notre groupe en janvier 2022, nous avions d'ailleurs pu établir le bilan du quinquennat qui s'achever marquée par la hausse des prix de l'immobilier et du foncier ainsi que par la baisse du nombre de nouveaux logements. Cette proposition de loi a donc un objet louable car elle vise, je cite, à renforcer l'action des collectivités territoriales en matière de politique du logement. Néanmoins, ce titre est excessif puisque cette proposition de loi ne concerne en réalité que les régions. Ne et ne porte que sur les résidences secondaires et ne consiste au final qu'à créer une nouvelle taxe. Le dispositif proposé n'apparaît donc pas satisfaisante pour 2 raisons principales, premièrement la création d'une nouvelle taxe régionale sur les résidences secondaires n'apparaît pas utile, alors que la possibilité donnée aux maires d'agir sur la fiscalité des résidences secondaires vient d'être renforcée. En effet, un débat sur la taxation des résidences secondaires, a déjà eu lieu au Sénat il y a à peine un mois lors de l'examen du projet de loi de finances 2023. Notre collègue Jean-François Husson, avait bien noté que la proposition du gouvernement d'élargir les zones où les communes sont autorisés à majorer de 60% la taxe habitation des résidences secondaires n'était que la suite de la réforme, je cite, non financée et bâclée de la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale. Finalement, dans un esprit de compromis, l'action notre groupe a choisi de doter de donner aux communes la possibilité d'augmenter la taxe habitation dans la limite de 25% sur les résidences secondaires sans augmenter la taxe sur le foncier bâti. Si nous ne sommes pas favorables à la création automatique, une nouvelle taxe. C'est aussi parce que parce que l'augmentation de la fiscalité sur les actifs immobiliers ne produit pas les effets escomptés. La délégation aux collectivités territoriales du Sénat l'a clairement démontré dans un rapport de mai 2020 relatifs aux communes face à l'inflation des prix de l'immobilier. Plusieurs dispositifs juridiques récents qui ont cherché à limiter l'augmentation du prix de l'immobilier par l'augmentation de la pression fiscale n'a eu que des conséquences marginal. Pire, l'augmentation de la pression fiscale a suivi la courbe de l'augmentation des prix. ce type de mesure ne peut donc pas être une situation à la crise du logement. Deuxièmement, le dispositif proposé ne vise pas les chefs d'actions pertinentes sur le terrain, nous pouvons le constater le problème du logement est avant tout un problème communal ou intercommunal en ce sens, ce sont les communes éventuellement les intercommunalités qui développent les politiques locales de l'habitat, par différents moyens, notamment les plans locaux d'urbanisme. Si la décentralisation a accru la complexité de la répartition des compétences de la politique du logement et de l'habitat. Avec les départements et les régions. Il n'est pas utile de renforcer cette complexité. Au contraire, il faut de la clarté. Les maires ne doivent pas être tributaire d'intervention extérieure. D'autres collectivités qui viendrait limiter aux contrer leur action d'autant plus dans un marché de l'immobilier où sont déjà présents. De nombreux acteurs privés. Ce constat est encore plus d'une nécessité dans les communes rurales qui représente de 88% des communes et 33% de la population et qui sont peut être l'une des réponses à la crise du logement. Je note ainsi que depuis la crise du Covid-19, les atouts des communes rurales sont plus reconnus et conduise à un changement de la mobilité résidentielle, un rapport de l'Insee publiée en décembre 2022 le confirme le souhait de migrer vers des communes rurales à augmenter depuis la pandémie. Enfin, chers collègues, en janvier 2023. Il n'est pas possible de débattre. La situation du logement sans évoquer. La mise en oeuvre Dusan. Cet objectif oblige à concilier les objectifs des politiques de l'urbanisme, de l'habitat et du logement avec de nouvelles contraintes. La sobriété foncière qui s'impose est une opportunité pour se saisir de certains leviers pour aménager l'habitat avait la densification des zones construites et la réhabilitation du bâti des centre-bourg y compris dans les espaces ruraux. Pour cela le fond Vert qui reprend. En partie le fond Free doit perdurer au-delà de de l'année pour laquelle il a été mis en place, ce sont des concentrés à la main des préfets favorise l'arrêt au propre, la réappropriation du bâti existant. Dans cette perspective, l'importance de ce du rôle planificateur des mères sera renforcée par la nécessité de penser et de mettre en oeuvre un développement équilibré à l'échelle de la commune vous le, vous l'aurez compris, notre groupe suivra l'avis réservé du rapporteur de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. L'accès à l'immobilier est devenu l'une des principales préoccupations de nos compatriotes. Et pour cause, le logement est désormais le 1er poste de coûts dans le budget des ménages. Ceci s'explique pardon dans par la hausse massive et généralisée des prix de l'immobilier depuis le début des années 2000, l'indice des prix brut des logements neufs et anciens a augmenté de plus de 180%. outre plusieurs mesures de la loi résilience climat adoptée en 2021 risque de compliquer la donne. Des interdictions de louer et de vendre des passoires énergétiques vont contraindre l'offre de logements disponibles et donc augmenter les prix. Ces mesures répondent à des objectifs environnementaux que nous partageons tous. Mais ces objectifs ne doivent pas nous conduire à ignorer la situation. De même, l'objectif de zéro artificialisation nette que nous partageons aussi limite considérablement les capacités des collectivités à recourir à l'étalement urbain, pour augmenter l'offre de logements disponibles, là encore les conséquences sur le marché de l'immobilier ne seront pas négligeables. Dans ce contexte national complexe certaines situations locales s'avère encore plus complexe. C'est notamment le cas des zones tendues ou le développement des résidences secondaires contrainte encore davantage l'offre de logement disponible pour les habitants de ces villes là encore nous avons tous conscience que ce phénomène concerne de nombreuses communes françaises créant ça et là des tensions entre la population locale et des habitants saisonniers. Nous pouvons donc nous accorder sur le constat mais diverger sur l'analyse des causes. En l'espèce le diagnostic selon lequel l'augmentation des prix de l'immobilier seraient dus aux résidences secondaires me semble spécieux. L'étude de l'Insee sur laquelle se fonde l'exposé des motifs preuve révèle 2 autres réalités qu'il serait malvenu d'ignorer. La première c'est la modification des structures familiales. Et avec elle d'augmentation de la proportion des foyers au sein de la population. Ainsi depuis 1982, le nombre de résidences principales s'est accrue de plus de 50%. Alors que la population n'a augmenté que de 20% sur la même période. Il y a donc aujourd'hui plus de résidence principale pour la population générale globale qu'il n'y en avait il y a 40 ans. La seconde réalité c'est que les résidences secondaires ne représente que 10% du parc de logements. Au cours des 20 dernières années, leur nombre n'a augmenté que de 35% alors même que l'comme je l'avais a rappelé à l'instant. Les prunes, les prix de l'immobilier ont augmenté sur cette même période de plus de 180% l'augmentation du nombre de résidences secondaires n'explique pas la hausse des prix généralisée de l'immobilier. Il m'a semblé important de rappeler ces éléments car ils expliquent pourquoi notre groupe ne soutiendra pas ce texte. Bien sûr, nous sommes favorables à l'objectif affiché à savoir renforcer l'action des collectivités territoriales en matière de politique de logements. Mais la proposition de loi que nous allons examiner se résume en fait à la création de taxes supplémentaires sur les résidences secondaires. S'il suffisait de taxer davantage les Français pour faire baisser les prix de l'immobilier, alors il n'y aurait pas de problème d'accès au logement en France. Car il faut le rappeler nous sommes le pays de l'OCDE où le poids des prélèvements obligatoires et le plus important après le Danemark. Enfin, le dispositif proposé risque de gêner les élus locaux. Anne effet il confie aux régions la possibilité de créer une taxe alors qu'il s'agit pour l'instant de décisions prises par les couleurs et les intercommunalités. Je termine Monsieur le Président qui demeurent les collectivités de proximité, cette taxe ne s'appliquerait. Outre qu'en zone tendue tendue lorsqu'elles sont déterminées par décret ce texte apporte donc une mauvaise solution à un vrai problème de société.

Quand Jean Ferrat chantait ses mots, il parlait d'une société moderne, que les jeunes quittaient un à un pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Aujourd'hui, nous vivons l'inverse, les jeunes veulent vivre au pays. Aucune région n'est épargnée par le fait qu'ils ne peuvent plus y vivre. La hausse des prix de l'immobilier du Foncier la multiplication des Herbiers NBA et des résidences secondaires oblige les jeunes et les catégories moyennes et modestes, à se loger toujours plus loin c'est une ségrégation sociale et spatiale qui se développe à grande vitesse Nous venons de l'entendre, est partagé sur tous les bancs et la volonté d'agir aussi la proposition de loi que mon collègue Ronan Dantec présente pour notre groupe monde que nous pourrions agir modestement mais commencer à agir sur deux niveaux, le premier niveau, l'effet de l'accroissement du nombre de résidences secondaires sur le prix de l'immobilier et deuxièmement la maîtrise foncière des villes et des métropoles, ce serait un 1er pas qui sera nous n'en doutons pas poursuivi, amplifié car il le faut et notre assemblée face à Air bien une bise et à la spéculation foncière saura se saisir de cette situation et nous l'accompagnerons dans ses propositions. Mais cette proposition de loi ne vient pas ici par hasard elle répond à de nombreuses interpellations de maires de communes littorales et touristique qui toutes et tous, sans la moindre exception dénoncent les conséquences directes et je vais citer ici les propos d'un appel que j'ai reçu du Collectif des maires du Val de Saire. Réduction de la population permanente de communes accélération du vieillissement fermetures de commerces et de services publics de classes voire d'école disparition des services médicaux et paramédicaux. Le premier article suscite des interrogations, voire des inquiétudes nous l'entendons. Sur la place des régions dans cette politique. Si cet article n'obtient pas un consensus. En revanche, l'amendement de notre collègue qu'Isabelle briquet qui propose de remplacer cet article par celui que nous avions voté collectivement pour décoléré des. des. Taxe foncière et es hrs répondrait aux inquiétudes venues des élus du Pays basque de Corse, de Bretagne, de Normandie, des Alpes ou des Pyrénées. Sans parler de ceux des métropoles. Si je commence la liste je ne la finirait pas car ce phénomène touche tous nos territoires cet amendement que nous avions voté très largement dans notre chambre a été, je le rappelle, supprimée par le 49.3. Nous pouvons donc rétablir cette disposition et donner un nouveau signal aux collectivités territoriales qui nous font confiance, de la volonté du Sénat d'être à leurs côtés. il existe des désaccords sur le premier article bien que nous pensions que les régions aient un rôle à jouer sur le deuxième, il ne devrait pas y en avoir les EPFL nous sollicitent et nous demandent des moyens accrus faite aux sénateurs d'outiller les territoires en renforçant leur pouvoir d'agir, devrait obtenir un consensus très large sur ces bancs. À moins les les EPFL en ont besoin, ils nous l'ont écrit. Évidemment, il pourrait y avoir d'autres dispositifs. Monsieur le Ministre, vous pourriez choisir d'augmenter les dotations à ces établissements publics fonciers pour les aider dans leurs travaux. Nous ne sommes pas persuadés que ce sera la voie choisie dans un temps court, c'est la raison pour laquelle nous disons donnons même à nos collègues les EPFL sont dirigées par les élus territoriaux donnons même à nos collègues la possibilité de choisir, comment il veut agir, et s'ils veulent agir avec plus d'autonomie fiscale. De ses structures et ses institutions aucune obligation mais un pouvoir de décider d'agir pour les collectivités territoriales de nouvelles marges de manoeuvre plus de pouvoir aux collectivités, ce serait finalement une décision magnifique de notre assemblée. Face à ce problème, que tout le monde constate. Merci cher collègue. La parole est à madame Nicole Duranton pour le groupe RDPI pour 4 minutes. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre. Monsieur le rapporteur, chers collègues. Commande exposée dans l'Expo comme énoncés dans l'exposé des motifs. Nous en avons tous fait le constat dans nos territoires respectifs depuis l'an 2000, la France a connu une hausse vertigineuse du prix de l'immobilier. Cette hausse a obligé les populations locales à se loger toujours plus loin de leur lieu de travail et de socialisation littoraux zone frontalière montagne grande ville est désormais certaines communes rurales, aucun espace n'est épargné. Mais l'augmentation du volume des résidences secondaires représentant aujourd'hui un logement sur 10 selon l'Insee n'est pas l'unique facteur déterminant. Cette hausse non il n'est pas exact de dire que tous les jeunes souhaitent rester dans leur commune d'origine. Bien au contraire, il est très sain pour un jeune est également pour un moins jeune de vouloir quitter à un moment ou un autre, sa commune découvrir d'autres horizons, d'autres environnements pour mieux y revenir plus tard. Les élus locaux trouve tout de même Avantage à la présence de ces résidences secondaires résidents qui n'ont d'ailleurs de secondaire que le nom, car beaucoup d'entre eux participent activement au dynamisme du territoire et au développement de la fameuse attractivité économique que l'on recherche temps. À titre d'exemple, dans les années 1960 1970. Mon père était adjoint au maire de ma commune en Normandie où la municipalité se réjouissait de l'engouement des Parisiens venant acheter à 150 kilomètres de Paris, des longères ou des vieilles fermes à retaper pour en faire des résidences secondaires il participait activement à l'entretien du Patrimoine bâti de la commune et en faisait d'ailleurs souvent leur retraite venu une résidence principale. Vous nous proposez d'employer une sur-imposition dans un objectif de réorganisation du marché local du logement pour tenter de dissuader les propriétaires de conserver des résidences secondaires. Je vous rappelle que nous avons voté au PLF dernier un élargissement de la disposition qui autorise les municipalités classé en zone tendue à voté une surtaxe à la taxe d'habitation pour les logements secondaires. Je crois qu'il nous faut conserver cet équilibre

peu juste et peu conforme à l'objectif que vous poursuivez. Le rapporteur a eu l'occasion de le rappeler dans l'article 1er, les régions ne sont pas à l'échelon pertinent pour mettre en place une nouvelle surtaxe, ce d'autant qu'elles ne sont même pas demandeuse de cette nouvelle ressource dans le second, la même logique est employé au profit des établissements publics 106 foncier pour financer la fameuse préemptions avec ses double augmentation de la taxe d'habitation on créerait un régime quasiment confiscatoire pour des propriétaires qui parfois ont simplement héritiers d'un bien familial qui qu'ils se sont engagés moralement à garder sans être pour autant la caricature du grand routier. En l'état cette PPL a été examiné par la commission des finances. Réuni le 25 janvier sur le rapport de monsieur Jean Baptiste blanc que je félicite, elle n'a pas adopté. Elle n'a pas été adopté en commission. Ce qui est un signal négatif très fort. Le groupe socialiste proposent sert de réécrire le premier Arctique pour décoléré la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la taxe foncière sur les propriétés bâties, quoi que plus consensuel, je ne pense pas que cette rédaction amendée serait de nature à améliorer l'état de droit. La corrélation des taux lorsqu'elle fut instituée n'était pas une lubie jacobine mais une mesure d'équité moins représentées dans les décisions municipales. Les propriétaires de résidences secondaires, fatigue s'acquitte pardon de la taxe foncière, au même titre que leurs voisins résidents permanents tout en niant pour pourtant moins recours aux services publics locaux. Pourtant si la taxe d'habitation a été supprimée pour les seconds, elle demeure pour les premiers, n'allons pas trop loin dans la surenchère. La justice fiscale. Oui, le racket fiscal. Non je mesure toutefois d'un certain nombre de. Je souhaite que nous puissions y travailler donc à l'avenir. Mais cette proposition de loi ne répond en aucun cas à ce problème. Raison pour laquelle notre groupe votera en large majorité contre cet été. Dans la suite de la discussion, la parole est à Isabelle briquet pour le groupe socialiste, écologiste républicains pour six minutes. Monsieur le président, Monsieur le ministre, hein. Monsieur le rapporteur. Monsieur le président de la commission des finances. Mes chers collègues. Cette proposition de loi portée par nos collègues du groupe écologiste solidarité et territoires traduit, nous l'avons vu un réel besoin pour nos concitoyens. Lutter contre la hausse des prix immobiliers pour garantir l'accès au logement à toutes et tous. qui est à la croisée des chemins de l'aménagement du territoire et la justice sociale appelle une véritables réponses politiques de lutte contre les inégalités sociales et la fracture territoriale. Mes chers collègues, à travers le logement. Il s'agit de garantir à tous les citoyens le droit de vivre mieux. L'inégalité face au logement accentue les autres inégalités sociales comme l'accès au travail à l'éducation aux soins aux loisirs. Nous devons donc engager les moyens nécessaires pour permettre d'abord aux ménages notamment aux plus jeunes ménages d'inviter dans leur bassin de vie près de leur travail, des écoles et des différents services publics et pour ce faire douter les communes des outils indispensables à la maîtrise de leur foncier et de leur tissu économique et social. Cette question du logement rentre également en résonance avec la perspective d'application du zéro artificialisation nette than qui nécessitent également un véritable accompagnement à destination des élus locaux. Avec les membres du groupe socialiste, nous partageons les objectifs affichés dans ce texte permettre aux citoyens qui le souhaitent de rester vivre au pays, comme on le dit familièrement. Nous proposerons donc trois amendements tendant à renforcer l'efficacité du dispositif. Ainsi, afin, donner un levier fiscal supplémentaire aux communes. Nous proposons la réécriture de l'article premier, tout en partageant les mêmes objectifs que l'article initial la décorrélation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de la taxe foncière sur les propriétés bâties nous semble en effet un moyen mieux adaptés aux besoins des collectivités. La situation actuelle de corrélation entre les 2 taxes n'est pas en effet sans conséquence pour les communes touristiques, lesquels voit la transformation des résidences principales en résidence secondaire entraînant un étiolement durable de l'activité sociale et économique. Nous souhaitons par cet amendement endiguer le phénomène continue d'accroissement des résidences secondaires au détriment des principales. Il permettra aussi aux communes d'agir plus librement sur le tour de la. Tout en contribuant à une prise de décision en adéquation avec les besoins locaux. C'est pourquoi, dans un souci de consensus sénatoriale cet amendement reprend la version présentée par le président bah lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2023, version qui avait été adopté très largement par notre assemblée. En effet si nous partageons l'objectif nous pouvons donc aisément nous entendre sur le moyen d'y parvenir. D'autant plus lorsque le moyen en question a déjà emporté l'adhésion de la majorité d'entre nous, surtout nos bon. Je ne doute pas que ce qui était pertinent, il y a quelques semaines le soit toujours aujourd'hui. Ce dispositif est une attente forte pour nombre de communes et je ne saurais comprendre que notre assemblée en décide différemment à l'occasion de la guerre de l'examen de ce texte, quand bien même serait-il porté par d'autres. L'éloignement. Des populations du à la hausse du coût des logements touche particulièrement les jeunes ménages. Elle a également un réel impact sur le tissu économique et social des collectivités où nombre d'habitations ont été convertis en résidences secondaires. Ce phénomène ne concerne pas uniquement les zones tendues, mais se développe également dans les zones moins denses qui voit s'aggraver le phénomène de dévitalisation de leur centre-, bourg. Nous proposerons donc un article additionnel visant à étendre la possibilité de majorer le plafond de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à toutes les communes qui le souhaitent. Ce dispositif ouvrira donc cette possibilité à toutes les communes impactées par ce phénomène de résidences secondaires. De même, nous étendrons la majoration possible de 60% aujourd'hui à 100% de la THG. L'article 2 de ce texte propose d'ouvrir une possibilité de taxation spécifique au bénéfice des établissements publics fonciers. Au regard de l'importance de leur mission. Ces derniers constituent de véritables outils d'aménagement du territoire et de maîtrise du foncier. Nous proposerons donc d'élargir le dispositif à l'ensemble des communes, afin d'en accroître la portée et d'en garantir une meilleure effectivité. En conclusion, cette proposition de loi. Le grand mérite de traiter un sujet primordial au coeur de la justice sociale est essentielle pour l'égalité des territoires. Les réponses apportées pourront certes être complétée néanmoins elle constitue une première avancée. Nous devons donc nous devons nous saisir pleinement de ces questions d'habitat et d'aménagement du territoire. C'est pourquoi le groupe socialiste, vous l'avez compris apportera son soutien à ce texte, je vous remercie. Merci cher collègue. Dans la suite de la discussion. La parole est à monsieur Pascal ça le veulent délit pour le groupe CRCE pour 4 minutes.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes, mes, mes chers collègues. Ça va sans dire que votre présence le ministre à la à la tout son sens. Parce que pour notre groupe. Il en va du devoir de l'état de, de garantir le droit au logement. Et la politique du logement. Je dirais pas qu'elle est abandonnée, mais elle est quand même assez relégué d'ailleurs avec des gouvernements successifs pas ce seulement le. Le vote. Je pense aussi à des actes législatifs hein moi j'étais pas là à ce moment-là mais je pense. Les dernières loi sur le logement notamment la loi Elan qu'ont mis quand même en difficulté les les bailleurs sociaux et ça a impacté le le logement social. Et évidemment le Patrimoine de ceux qui n'en ont pas, ça c'est évident. Certaines. Évolutions législatives n'ont pas permis de faire du droit au logement, une norme. Enfin je, je veux dire. Une norme un droit une une réalité pour tous nos citoyens et citoyennes et là tout le monde l'a évoquée depuis tout à l'heure, on a un rapport alarmant de la Fondation Abbé Pierre. On peut décliner dans nos, dans nos départements respectifs. Nous en Val-de-Marne, c'est des dizaines de milliers de demandeurs de logements. Vous voyez, on n'est pas sur une petite échelle de de périmètre de de de problèmes et on viendra bientôt, vous le savez on aurait dans allemand fin mars début avril à un état des lieux. Monsieur le Ministre, ou je pense vous serez attentif. C'est le bilan triennal de l'application de la loi SRU. Voilà. Je suis aussi dans un département, le Val-de-Marne. Où. Près d'un quart des villes ne respectent pas la loi SRU. Et donc vont être encore sanctionné par l'État.

Un petit retour sur le passé. Je me rappelle. Je n'étais pas ici mais il y avait la loi notre. Et là on n'a pas tous été d'accord, c'est le moins qu'on puisse dire parce que nous, nous avons voté contre la loi, l'autre qui était une nouvelle. Organisation territoriale de la République. Mes chers collègues et chers sorti un amendement du 20 janvier 2015 qui était porté par mon ami Christian Favier Madame Assassi Cukierman et l'ensemble des du groupe à l'époque qui demandait les auteurs de cet amendement souhaitait que la garantie du droit au logement décent et indépendant demeure une compétence de l'État. Donc voilà c'est ça c'est fondamental. Après ça fait débat. Nous réaffirmons nous en profitons, vous nous en ont donné l'occasion de réaffirmer que ça doit être la compétence. De l'État. alors après la on a des dispositifs qui nous sont proposées d'aide au départ. Mes collègues le savent, on allait s'abstenir. Pourquoi parce que nous sommes que la région n'était pas le périmètre dans appui un périmètre opérationnel. La région n'a pas cette compétence. Dans la projet de loi qui nous était proposé c'était optionnelle c'est normal puisque la libre administration des collectivités. Donc les régions la recette de cette 2ème taxe sur les en secondaire mais n'aurait pas eu l'obligation de la fête au logement, la possibilité donc il y avait beaucoup de limites quand même sur cette affaire et donc. L'intention était louable mais la modalité était pas efficace. Là on a un amendement qui renvoie la question de la décorrélation taxe d'habitation, taxe foncière qui le renvoie aux communes. Donc c'est un autre projet de loi. Qui est plus conforme à ce que nous pensons, pensons que notamment la commune et les départements sont les 2 leviers essentiels. Aux côtés de l'État aux côtés de l'État pour qu'on réponde aux questions des logements c'est des lois. Ça fait plaisir de voir que le débat parlementaire. Il peut être passionnant parce que des fois on n'a pas que des fans Renault savoir d'un côté ou de l'autre de l'hémicycle, c'est qu'à un moment où on travaille et puis on essaye de trouver des solutions, donc je vous le dis, nous on était sur une position d'abstention on aurait voté l'article de. Ça je l'avais dit en commission des finances, là on votera l'amendement que que Isabelle Bris qui a. Expliqué qu'elle va encore mieux expliquer tout à l'heure et ce qui nous amènera à voter favorablement à ce projet de loi. Avec limites La parole est à monsieur Jean Michel Arnaud pour le groupe Union centriste pour six minutes. Il à monsieur le président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous avons donc à examiner ce texte proposé par Ronan Dantec, notre collègue. J'en profite pour saluer le travail réalisé par. Notre rapporteur Jean-Baptiste Blanc. La politique du logement, vous le savez pas nouvelle. Occupe une grande partie de de nos travaux. Le fait d'être logés surtout logés dans des conditions décentes, est un élément. Non seulement structurant pour toute démarche individuelle mais également un élément de cohésion sociale majeure pour notre pays. Pour autant, notre pays fait face à un manque de logements dans les faits, nous avons à faire à un déséquilibre structurel entre l'offre et la demande. Et notamment dans les zones touristiques montagne littoral le développement des résidences secondaires accroît les tensions sur ce marché. Je le vois dans mon département les Hautes-Alpes ou la déconnexion entre le prix d'immobilier. La réalité du marché entraîne des difficultés grandissantes pour les jeunes populations mais aussi parfois pour des élus. J'ai en tête un maire d'une des stations des communes de station de Serre-Chevalier. Qui ne peut pas être propriétaire dans la propre commune qui dirige. Il n'est que locataire ne pouvant pas accéder au marché du logement. Dans ce contexte. La facilité effectivement d'avoir un débat récurrent ici dans notre assemblée. Sur le recours au levier fiscal. Et la présente proposition n'y déroge pas pour ce qui concerne les résidences secondaires. Depuis le 1er janvier 2023, vous le savez toutes et tous à la suite de la suppression regrettable de la taxe d'habitation. Pour les résidences principales. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires s'applique de manière générale à des locaux qui, sans être occupé en tant que résidence principale sont meublé. Et propre à l'habitation cela les distingue aussi bien des résidences principales que des logements vacants. Je pense qu'il serait utile ultérieurement que notre assemblée se penche aussi sur les conditions d'accompagnement fiscal de ces résidences meublées et une des idées soumises notamment par des élus de la montagne serait de veiller à ce que les multipropriétaires de logements meublés soient dans l'obligation de louer une partie de leur Patrimoine en résidence principale pour avoir un effet de levier sans pour autant pénaliser l'attractivité que peuvent avoir nos résidences secondaires dans nos zones touristiques. L'exposé des motifs de la PPL précise qu'il s'agit d'un outil de reconquête de l'habitat en France. Belle ambition cette volonté politique à laquelle notre groupe souscrit naturellement est louable. Toutefois les 2 articles de cette proposition de loi ne sont pas apporter une réponse adéquate, un problème dans l'étendue ne saurait se limiter aux résidents secondaires. Tout d'abord cela a été rappelé, il est proposé de créer de taxe additionnelle à la taxe d'habitation dont une serait instituée au profit de la région. L'objectif serait d'accroître les marges de manoeuvre du conseil régional à la conduite, sa politique, la maison de territoire, notamment au titre des établissements publics fonciers locaux et régionaux. L'échelon régional n'est pourtant et on le vit tous dans le cas de nos expériences municipales passées ou actuelles n'est pas le plus pertinent sur la question des logements. Dans les territoires et de manière opérationnelle sur nos territoires, bien que les conseils régionaux disposent de la compétence pour promouvoir le soutien, l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat. Ils n'ont que peu investi dans tous les cas dans ma région ce Champ qui relève historiquement du niveau communal et intercommunal. À noter d'ailleurs que, une grande partie des régions ça été rappelé tout à l'heure par le rapporteur ne sont pas forcément demandeuses en la matière pour pouvoir restaurer une nouvelle fiscalité en la matière. Aussi le caractère facultatif, cette taxe additionnelle pose un problème. Si le cas échéant certaines régions l'appliquer et que d'autres y renoncer, on assisterait à une concurrence fiscale. Difficile. Apprécier avec des disparités entre les différents territoires. C'est pourquoi la taxation des résidences secondaires doit s'apprécier en fonction des territoires et des circonstances locales au sein même non départements il y a des communes, avec un nombre de résidences secondaires faible voire inexistant et dans le même temps des communes touristiques dans le taux de résidences secondaires dépasse les 70% de tous les logements. Je rappelle aussi que la TH RS demeure une source de revenus pour le bloc communal. Cela est particulièrement effectif depuis la possibilité pour les communes situées dans les zones géographiques définies par l'article 232 du code général des impôts de majorer leur part. le revenant de Th RS d'un pourcentage compris entre 5 et 60%. J'apprécie également les propos rassurants de Monsieur le Ministre tout à l'heure dans son introduction, nous laissant entendre que, dès 2024, cette taxe pourrait être effectivement mobilisées avec des délibérations à prendre pour nos collectivités avant octobre de cette année. En parlant de cette possibilité de majoration. Un autre élément mis en exergue par le rapporteur a également retenu mon attention. Le risque d'inconstitutionnalité des mesures proposées. Dans l'hypothèse où le conseil régional et l'établissement plus foncier fixerait le taux des de taxes prévues par la présente proposition taux maximum de 25% le taux de taxe d'habitation résultant de l'application de la proposition de loi, sur un total de 86% de la valeur locative dans une telle situation. Le juge constitutionnel ou administratif pourrait considérer cette imposition comme confiscatoire en violation du principe d'égalité devant les charges publiques. Vous l'avez compris, mes chers collègues, le groupe Union centriste votera contre cette proposition de loi n'appelle le ses voeux un traitement global. La problématique du logement. Accès à la propriété. Lits froids chaud évidemment, construction de logements sociaux. Les sujets ne manquent pas. Le futur examen de la proposition de loi visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de. Zéro artificialisation nette au coeur des territoires sera certainement l'occasion d'aborder en profondeur ces dossiers tant sur le point de vue fiscal que du point de vue réglementaire, je pense en effet qu'il est absolument indispensable de reterritorialisation les objectifs de réduction de l'artisanat et son aide de sol. Je crois qu'il est également proposée par un certain nombre de nos associations. Le fait de conserver pour certaines communes, notamment les plus rurales un droit minimal de constructibilité par commune. clair. Monsieur le ministre et que le gouvernement écoutera et entendra ses propositions car elle dépend aussi d'une politique d'aménagement du territoire et de développement de logements à due proportion au moins équilibré dans nos territoires entre les zones rurales et les zones urbaines. Je vous remercie. Merci cher collègue. La parole est à monsieur Max Brisson. Pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Monsieur le président de ce ministre ne se de rapporteurs, mes chers collègues, je le dis es prise à présent je partage le constat que dresse cette proposition de loi présentée par Ronan Dantec. Il est primordial d'un effet d'agir pour aider les collectivités locales à contenir les excès de la transformation accélérée de l'habitat dans certaines zones tendues. Ainsi, dans mon département au Pays basque, il faudrait qu'Espagnac et puis CP pour dire la même chose. La part des résidences secondaires représentent désormais 15% du nombre total des logements et près de la moitié dans certaines communes du littoral 900 résidences secondaires apparaissent chaque année dont 600 était auparavant habiter de manière permanente. Cela produit une récente et spectaculaire raréfaction de l'offre de logements en location durable et une dangereuse crise du logement aux ramifications politiques préoccupante. Cette croissance exponentielle des résidents secondaires s'appuie sur celle des locations saisonnières qui permettent aux acheteurs des premières d'intégrer le rapport des secondes dans leur montage financier. Les conséquences sont alarmantes. La flambée des prix de l'immobilier. L'envolée des loyers à l'année la multiplication des locations précaires souvent illégale sur 10 mois pour libérer les logements aux beaux jours cette spirale infernale éloigner les ménages toujours plus loin des centres urbains. Ses premières victimes sont les jeunes, les personnes les plus fragiles, les plus isolés, les étudiants, les apprentis les familles modestes. Dans ce contexte, les 21 communes basques classés en zone tendue ont depuis plusieurs années déjà mis en place la procédure de changement d'usage et la majoration maximale de 60% du taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et partout appliqué et ceci indépendamment des sensibilités politiques des municipalités. Cela n'a pas suffi. Voilà pourquoi la communauté d'agglomération du Pays basque y'expérimenté et expérimentera dès le 1er mars. Un système de compensation obligeant pour tout bien dit sur le marché de location saisonnière à mettre un bien nouveau sur le marché à l'année. La mesure est drastique pour autant résorbera-t-elle la crise du logement. Je ne le crois pas, cette crise est bien global et complexe épouse les élus de tous bords à chercher des solutions dans ce cadre, cette proposition de loi propose de taxer au profit des régions et des EPFL j'en conviens, il est toujours alléchant de créer une taxe additionnelle il va en attribuer des bénéfices aux collectivités territoriales. Je ne doute pas qu'elles en feront bon usage et je reconnais que la PPL pose le sujet mais raisonnons nous si l'issue de cette crise était uniquement la création de taxes supplémentaires. Je crois qu'elle aurait été et Isabelle aisément résolu, même si cher rapporteur le besoin de recettes existe et je suis convaincu que la réponse passe d'abord par la production de logements locatifs aidés et d'accession sociale à la propriété. Or, et particulièrement dans ces territoires. Au-delà de la raréfaction du foncier de son prix. La production devient insoutenable pour les bailleurs sociaux à la fois affaibli par l'augmentation des coûts des matériaux de construction et par la réduction de leurs fonds propres. À force de leur avons fait les poches. Ceux-ci sont confrontés à l'inflation, confrontés à l'inflation non plus la capacité d'assurer l'équilibre des opérations dans ces territoires ne nous foot il tombe pas chercher un nouveau modèle de financement du logement social dit il va également poser le sujet des zonages et des plafonds d'accès au béret c'est au Berry pour apporter une réponse à la part des classes moyennes qui ne peuvent plus accéder et qui se trouve peu à peu évincé de ces territoires ne sont-elles pas aussi devant nous les questions visant les avantages fiscaux dont bénéficient encore les locations saisonnières, par rapport. Location à l'année et que le gouvernement a conservé malgré nos votes dans cette assemblée, par le 49.3. La limite du nombre de jours de location saisonnière autorisé pour les résidences secondaires d'une résidence principale ou résidence secondaire est également un sujet explorer la procédure de changement d'usage qui ne devrait plus être une simple formalité mais s'appuyer sur un véritable agrément pour donner la main aux maires en leur permettant d'exercer un réel contrôle contrôle est une piste également explorer n'est-ce pas là quelques pistes en effet qui finalement renvoient à la responsabilité de l'État qui dans ces territoires devraient être animateur et stratège et non prescripteurs permanent de normes et censeur impitoyable. C'est à lui de rétablir les conditions qui permettront de relancer la construction de créer une offre équilibrée de logements locatifs et un qui sont sociale à la propriété et en fin de restaurer des parcours résidentiels

Merci monsieur le président, ainsi que cela a été dit tout à l'heure donc cet amendement vise à réécrire intégralement le premier article de la proposition de loi pour proposer un dispositif ayant un objet similaire mais qui serait son contexte plus plus efficace et si j'en j'en juge les hein. Les interventions qui ont été faites précédemment, il a, il m'a eu l'air de convaincre, pas mal de monde sur les différents bancs il vise en effet à modifier l'article 1636 bé sexy du code général des impôts afin de décorer les la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la taxe foncière

Présentée par le président bah lors de l'examen du projet de loi de finances hein qui est qui est vraiment reprise. Version que nous avions communément. À ce moment-là. Donc la la corrélation comme j'ai pu le dire aussi tout à l'heure entre. La TA Giresse et et la taxe sur le foncier bâti. N'est pas en effet sans incident hein néfaste pour les communes touristiques C'est pourquoi ce. Cet cet amendement me paraît pleinement pleinement justifiée. Cette adoption permettrait aux communes d'agir plus librement sur le montant de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, tout en contribuant à une prise de décision davantage en adéquation avec les besoins locaux puisque c'est bien de ça. Dont il s'agit et où, pour beaucoup, nous aussi hein. L'échelon régional ne semblait pas pertinent de ce fait, donc là on est vraiment au plus près des des territoires et des besoins locaux.

Une chose qui qui qui m'interroge relatives à cet amendement, c'est le caractère un petit peu étranger à l'article 1er de la PPL, c'est-à-dire que le, l'article 1er. Invoque bien la création d'une taxe additionnelle à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Et quand on lit l'explication dans les motifs aux fins de financer de l'ingénierie dans le cas de la politique du logement et on parle de Anne je le 18 mai, c'est un peu l'esprit. Là vous proposer tout à fait autre chose. On de renforcer le bloc communal. Je trouve que c'est un petit peu étranger au Cadre posé strictement par l'article 1er néanmoins. Si je trouve toujours comme mes collègues. La la question fort légitimes et extrêmement fondé et qui appelle à être traiter à un moment donné, notre histoire. Ça n'empêche que elle est un petit peu prématuré à mon sens, eu égard aux travaux actuels du Sénat il y Dan PPL than qui arrive, on ne sait pas strictement le logement mais Lausanne va permettre de traiter beaucoup de politiques publiques en même temps au sein de cette PPL cette PPL c'est au mois de mars. Ensuite en ce qui concerne la commission des finances et je salue mon président. Il y a une mission de contrôle sur les EPL. Qui va être déclenchée dans les prochaines semaines. Donc on va. Voir ensemble, si les les EPL sont vraiment armée et suffisamment musclé pour appréhender le foncier dans le cadre, tous ces sujets qui se posent à nous logement than. Et autres, donc cette mission va commencer. Par ailleurs le format n'est pas encore établi, mais il va y a bien, il va bien avoir une suite. À la mission conjointe de contrôle sur Lausanne qui sera le financement et la fiscalité Dusan ou souvenez qu'on a déjà rendu un rapport ensemble à la commission des finances. On a saisi le Conseil des prélèvements obligatoires sur le sujet qui fait des propositions cette matière là qu'il va falloir travailler. On est tous d'accord oh je reprendrais volontiers les mots. De Ronan Dantec, nouvelle mission nouveau financement non mais voilà on est tous d'accord sur le, l'objectif, c'est-à-dire qu'il va falloir inventer là des fiscalité locale verte pour appréhender le foncier et au-delà. Lausanne en ce sens cette PPL est un peu prématurée compte tenu des travaux qui qui nous attendent qu'on va faire ensemble. Après, permettez-moi. Au-delà de ce qui allait encore 2 arguments. Le 1er qui est celui de la hausse potentielle de la fiscalité locale, c'est aussi une réalité et le second c'est que il a été voté des dispositions au sein de la loi de finances, le ministre-, là, là les a rappelé. Dans ces dispositions. Il faut qu'on voie si ce que ça donne, si elles sont opérantes. Ou pas vraiment. Je rappelle l'article 73 par exemple pas étendu le périmètre d'application sur la taxe sur les logements vacants à l'article 74 à à augmenter le taux de la taxe sur les logements vacants en le faisant passer de 12 et demi à 17% la première année et 25 à 34%. La seconde année, donc ça va dans le sens du présent amendement. Et il semble donc important de laisser un peu de recul pour voir si tout ça fonctionne pas comme le, comme je vous le disais donc pour tous ces arguments et en l'état de la discussion. Je formulerai un avis de de de retrait. c'est pas une proposition de loi sur les résidences secondaires même si beaucoup d'interventions ont été centré sur la question des résidences secondaires. Donc et ben il me semble que l'amendement de Madame correspond totalement libellé de la loi, donc il n'est pas du tout. En dehors de nos préoccupations. Nous avons mis les régions. Dans la boucle d'abord parce que la loi note leur a bien donné une compétence en la matière. Il est vrai qu'elle l'utilise de manière différente. Il est vrai que l'arrivée des méga-régions. Qui n'était pas prévu dans le l'esprit initial de la loi notre rend aussi les choses plus difficiles sur le terrain Nous allons payer très, très longuement les errements de Manuel Valls sur ce point mais très clairement. Les régions vont devoir de plus en plus intervenir sur la question du logement sans aménagement du territoire sans équilibre de l'emploi. Nous n'y arriverons pas. Donc, le sens de l'histoire, c'est l'arrivée de plus en plus forte des régions sur cette question et avec leur puissance. Économique, donc c'était le sens de notre amendement, il est faux de dire que les régions n'en veulent pas. Certaines régions n'en veulent pas, ils nous avions bien prévu quelque chose d'optionnel. Effectivement, nous restons. Par rapport à mon camarade communiste des régionalistes. C'est une différence. D'analyse politique mais la région viendra ça j'en suis absolument convaincu. On attendant sur cette proposition de Madame. Que nous allons voter. Il s'agit simplement de rétablir ce que le Sénat a déjà voté très largement. Alors monsieur le rapporteur, essayer de trouver un argumentaire pour que politiquement, finalement ça ne reviennent pas Un, un groupe de la minorité puisque c'est ça mais je pense que vraiment on a besoin de revoter cet amendement. La question de la décorrélation est absolument centrale. Le 49.3 non démocratique a empêché que notre proposition votée par le Sénat soit discuté donc nous passons dans l'urgence par une proposition de loi pour remettre ça, il faut construire sur ma collègue donc effectivement je pense qu'on devrait retrouver le même consensus que lors du débat initial. Merci Madame Espagnac. Oui, monsieur le président. Merci, sur la suite de monsieur Dantec je voudrais moi aussi soutenir complètement cet amendement en proposant la réécriture de l'article de loi, c'est une occasion pour nous tous d'apporter une réponse consensuelle et efficace à un problème qui frappe de plein fouet de tri de de nombreux départements en particulier mon département des Pyrénées-Atlantiques mais mais comme tous les autres en Corse. En Bretagne, également. Rappelons-nous, rappelons-nous en effet que lors du budget déjà nous notre assemblée s'étaient accordés sur l'épineuse question de la décorrélation de ces de taxes lors de l'ESA bien du budget nous avions adopté à l'initiative de Philippe Bas comme cela avait été dit un amendement visant à permettre à compter de 2023. Une des liaisons entre le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties afin de donner davantage de morts de manoeuvre aux communes souhaitant utiliser ce levier fiscal pour lutter contre le phénomène de sous-, occupation des des Monsieur le rapporteur. J'entends et je fais moi-même partie de la commission Lausanne mais je crois qu'il y a urgence et je crois que ce sont deux choses aujourd'hui complètement différente, même si nous évoquerons le problème je pense qu'aujourd'hui, les communes sont en attente de décision rapide de notre part. Le gouvernement a dans l'élaboration du texte sur le. Il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49 3 de la Constitution préféré supprimer cette disposition et c'est une grande erreur, c'est une erreur car la décorrélation daté HRS et de TFPB que prévoit aujourd'hui le code général des impôts a une incidence majeure pour les communes touristiques leur fort potentiel touristique entraîne une conversion massive de nombreux logements en résidence secondaire. Les conséquences pour ces communes sont bien connus et implacable inflation des coûts de logement exode de la population locale en particulier des jeunes ménages n'ayant pas les moyens de s'y installer. Il nous faut donc être efficace et pragmatique sur cette question efficace en ce sens la décorer l'action entre la taxe d'habitation et la taxe sur le foncier bâti, est une solution adaptée pour lutter contre l'accroissement des résidences secondaires au détriment des résidences principales et contribuer à la revitalisation des communes concernées pragmatique et en ce sens afin d'éviter tout le 19 le pardon le dispositif proposé encadre cependant la décorrélation aussi l'adoption du présent d'amendement donnerait à nos communes la possibilité d'agir plus librement sur le montant de la taxe d'habitation soi-disant secondaire en fonction des besoins locaux. Merci. Mon intervention sera très complémentaire de celle de fêter Espagnac. Je comprends cher et Jean-Baptiste Blanc. Une partie de vos réserves mais seulement une partie de vos réserves. Quand vous nous dites c'est prématuré. Vous parlez comme Gabriel Attal lors du débat de sur le, la loi de finances 2023. Or il y a urgence comme Frédérique Espagnac Coupe d'une CMP. Moi je ne peux pas revenir dans mon territoire en disant c'est prématuré. On va faire un groupe de travail, moi je ne veux pas à porter ce discours là tellement la crise est prégnante et tellement la crise peut prendre de mer des répercussions sociales et politiques extrêmement grave. J'étais en colère lorsque le gouvernement après le 49.3 a fait disparaître mes amendement pourtant voté largement par cette assemblée et l'amendement de Philippe Bas. Je vais donc être cohérent. L'amendement briquet bah oh bah briquet comme on le veut et Monsieur bas pourrait demander des droits d'auteur mais vous avez donné ma chère collègue Opéra Copyright. Je l'ai soutenu, je l'ai défendu de loi. L'examen du projet de loi de finances et donc en cohérence. Je le voterai cette décorrélation qui n'est pas confiscatoire qui est à la marge cette décorrélation est nécessaire. Donnons aux communes les moi hier d'agir face à une situation de crise tous les mois. Hier, toutes les mesures seront bonnes. C'est dans un ensemble global, c'est pour cela que j'ai interpellé monsieur le midi tout à l'heure sous nos politiques plus globale, mais ne disons pas dans, à toutes les mesures parce que ça fait longtemps que l'on attend une disposition globale.

cependant moi non plus la la réponse ne me semble pas prématuré ce que cette décollera cette décorrélation et moi aussi je l'ai fait depuis le. Et. Est attendu d'une attente vraiment très très fort hein de de nombre de communes et en fait elle n'obère en rien. elle n'obère absolument pas aucune évolution future c'est c'est. Pour moi c'est un non sens de. De, d'amener cet cet argument-là. C'est bien un dispositif qui pourrait ça s'appliquer pleinement et qui rendrait grandement service un nombre de collectivités. Merci monsieur Calvet. Et moi je trouve que d'une part. Il y aura des dispositions qui ont été prévues dans la haute finance pour 2023 mais ne sera applicable qu'en 2024 et encore. Elle ne concerneront que les quelque 4000 communes qui auront pu être identifiés. Selon quels critères. Je ne sais pas. Mais identifiés comme étant des zones tendues. Or nous, nous nous apercevons clairement en Bretagne que les zones tendues, sont un peu partout donc il est urgent d'agir. Il est urgent que l'on dispose de leviers fiscaux tels que ceux qui ont été prévues dans la loi de finances de prendre le 23. J'aimerais bien que l'approche, Monsieur le Ministre soit un peu élargi, parce que la réalité des difficultés. Elle est plus générale qu'on ne le pense hein et. Dans cet esprit, je trouve que l'idée de de d'écorner le taux des taxes est absolument nécessaire aussi parce que d'une part il faut. Laisser de la liberté aux élus locaux pour la gestion de la stratégie fiscale et puis d'autre part, il faut leur donner des outils pour pouvoir justement dégager des moyens permettant d'apporter des réponses aux logement et je pense que cet amendement va tout à fait dans ce sens. Donc moi je suis, je le voterai bien entendu parce que ça ça permettra d'avoir des outils pour cela. Ce bruit. monsieur le président. Chers collègues, monsieur le rapporteur, m'a fait remarquer tout à l'heure que dans, dans ma DG. J'ai fait un lapsus très significatif. J'ai en effet parler de décoller ration au lieu de décorrélation mais c'est qu'effectivement j'étais un peu en colère comme je pense beaucoup sur ces bancs en colère de voir que l'amendement bah briquet et j'ajoute Breuiller puisque j'avais déposé un amendement équivalent chers collègues que c'est-ce amendements que nous avions portée sur tous les bancs. Avait été rejetée par un 49.3 comme c'est hélas souvent le cas pour les mesures qui viennent soutenir les collectivités territoriales. Alors oui je veux reprendre ce lapsus pour dire qu'il y a un peu de colère mais qu'il y a surtout nécessité de déco relais. en décor l'an nous nous donnons à nouveau un signal au gouvernement qu'il est urgent d'agir, qu'il est nécessaire de faire les premiers pas et de reprendre que nous avons voté ici en loi de finances et cher Jean Baptiste blanc ça n'est pas prématuré de faire un 1er pas nous sommes certains que ce 1er pas n'est pas à la hauteur des enjeux dont nous parlons ici les uns et les autres et que nous mesurons dans nos territoires, nous savons très bien que cette proposition de loi que nous vous présentons ne réglera pas la totalité du problème que nous avons ici, évoquées et dont nous avons tous souligné la gravité mais il vaut mieux faire un 1er pas que rester en stand-by. Et donc pour ma part évidemment je voterai cet amendement et je nous invite à avoir un vote conforme à celui que nous avons eu en PLF. Oui, merci Monsieur. Le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je pense qu'on est, on prend tous conscience, chacun avec ses mots. De la portée. Et de là. Limite de la portée de la proposition de loi, on est honnête. Voilà moi je vais pas vous dire que cette loi-là va résoudre mais 93.000 demandeurs de logement sur l'exercice 2021 avec 7500 logements. Je vous le disais tout à l'heure j'ai dit communes carencées il y en a quatre ou l'État obligé de faire préemptions pour créer 131 logements donc j'ai, il faut avoir la mesure et de l'humilité. Néanmoins là on a un sujet. C'est pas un cavalier le le. L'amendement qui nous est proposé il réaffecte à un autre niveau de collectivité. Des moyens, on était au départ sur la région et là, on finit par cet amendement sur la commune. Donc j'ai plutôt tendance, je l'ai dit tout à l'heure à encourager encourager cet amendement sur la question des des travaux prématuré. Moi j'ai du mal à suivre. Je pense qu'il y a pas de Trévoux prématuré quand il y a débat dans l'hémicycle. Bah oui. C'est que forcément ce qu'on décide, est ce qu'on débat ici, fait des joies fait déjà un peu loi. Forcément, donc c'est utile. Donc je pense qu'on est pas dans une situation on peut utiliser cet argument de deux prématurés. Alors après je vous le dis tout de suite, ça nous fera gagner du temps sur tout à l'heure si cet article 1 est voté, je le souhaite vivement. Alors là nous voterons la projet de loi. Par contre, vous avez bien compris que s'il est pas voter. On revient au texte initial, et là il a affectation à la région et ce qui amènera notre groupe ça s'abstenir. Oui, on est dans un débat constructif. Merci Monsieur Merci monsieur le président. Je ne crois pas du tout qu'on soit. Dans un moment prématuré. Moi ça fait depuis mon élection, ici en 2017 que par des amendements. J'ai été un peu lanceurs d'alerte je pense sur la crise du logement et la question du développement excessif des résidences secondaires dans les zones très touristiques en l'occurrence Paris. Et des meublés touristiques. Répondu avec un peu d'indifférence parce que ça ne correspondait que ça ne répondait qu'un problème parisien. Mais ce problème parisien c'est aujourd'hui développer à toutes les autres zones touristiques, je pensais à la façade Atlantique à la Bretagne aux Pyrénées Atlantiques à la Corse et continuera de se développer. Il ne faut pas avoir des outils qui soit toujours en retard sur la crise du logement et il s'agit pas de stigmatiser les résidences secondaires, mais d'empêcher que leur développement deviennent un véritable problème pour l'accès au logement des habitants d'un territoire et ensuite pour tout le développement et la stabilité elles-mêmes du territoire donc ne refusons jamais un outil qui permet d'aller plus loin. Je sais que notamment. Collègue Brisson et Frédérique Espagnac avait. Fait adopter un amendement sur les meublés touristiques ici qui n'a pas été retenu dans le 49 3. C'est dommage parce que les outils que nous votons sont déjà tellement faible par rapport à l'ampleur de la crise du logement qu'il ne faut absolument pas s'en priver et montrer aussi notre volontarisme et notre notre détermination à apporter une réponse à un problème d'accès au logement qui va continuer de se développer et qui est un grand danger pour pour beaucoup de territoires de notre pays et plus seulement les métropole très attractive, et les des métropoles ou d'une ville comme Paris. Merci monsieur le président, mes chers collègues. Effectivement, la France est championne. Par rapport au taux de résidences secondaires. C'est pas ça le problème en soi puisque de nombreux Français aspirent à avoir une résidence secondaire mais on partage un constat sur tous ces bancs, c'est qu'il y a une problématique logement aujourd'hui, la situation n'est pas satisfaisante. On le constate. Je veux dire socialement, c'est profondément injuste. Lorsque l'on voit de jeunes actifs, qui sont obligés de faire des migrations quotidiennes pour aller sur leur lieu de travail. Je parle de la Bretagne en particulier sur les zones littorales. Mais on le trouve dans bien d'autres endroits c'est économiquement néfaste néfaste pour les entreprises avec justement une recherche pour loger. Les salariés qui est très difficile aujourd'hui et c'est écologiquement non soutenable. Avec toutes ces migrations pendulaires qui conduisent. À vraiment un gâchis d'énergie à de nombreuses pollutions donc on partage ce constat sur ces bancs. Je pense que le Sénat, une fois de plus, peut se grandir à avoir une position complètement transpartisane sur un amendement qui a déjà été voté. Nous sommes là clairement dans une démarche d'autonomie fiscale que nous défendons sur tous ces bancs. Et je pense que nous ne devons absolument de donner un signal dans chacun dans nos régions, dans nos départements face à ce problème qui est vraiment un problème qui se généralise, même à l'intérieur de région qui jusque là n'étaient pas soumis à cette pression. Moi je pense ah pimpon qui se trouve une commune dans mon département qui est loin du littoral et qui elle-même est soumise à cette pression. Oui merci. Je pense que nous apprécions tous le petit tour de passe-passe. 2 à nos amis du groupe socialiste pour nous mettre soi-disant en défaut, mais juste pour dire que la loi de finance c'est quand même la loi qui parle de la fiscalité et là, à vous entendre avec cet amendement on doit résoudre le problème de la politique du logement, le problème de la fiscalité locale. Le problème de l'autonomie fiscale des collectivités. Donc je pense qu'on est face à une multitude de problèmes en loi de finances, on a lancé des messages au gouvernement. Il nous a invités à participer à moultes groupe de travail on est désormais le 2 février, aucune invitation n'est arrivée jusqu'à nous et on vous a notamment parlé de ce sujet de la fiscalité locale et je pense que vous vous attaquez pas du tout au problème puisque vous-même dans le 49.3, vous avez décidé de reporter de 2 ans. Le début de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et je pense que l'injustice dont on parle ici sur les résidences secondaires. Elle se pose pour tous les Français sur la résidence principale avec des valeurs locatives qui sont complètement décorrélé aujourd'hui de la valeur vénale et de la valeur d'usage, donc il faut peut-être plus tôt que aujourd'hui voter cet amendement qui résout enfin qui traite d'un petit problème à défaut peut-être de savoir si le réseau de vraiment attaqué aujourd'hui le Champ de la fiscalité locale avec tous les qui ont été abordés aujourd'hui donc peut être nous changerons pas de pied mais en tout cas parce qu'on n'est pas du tout dans le même contexte, nous voterons contre aujourd'hui mais en tout cas nous maintenons qu'il y a urgence à s'attaquer à ce sujet de la fiscalité locale, dans sa globalité. Oui monsieur président. Je crois que le, le débat est effectivement des plus passionnants. Je je constate. Que sur le, l'amendement de Madame briqué. Cet amendement est largement partagée par les territoires qui dispose de résidences secondaires massivement. Que ce soit des territoires de montagne sur des territoires du littoral et nous ne pouvons pas être insensible à la possibilité pour les collectivités locales de pouvoir asseoir leur fiscalité sur les résidences secondaires de manière détachée de la fiscalité qui repose sur les résidents principaux donc à ce titre-là. Une majorité. De membres du groupe centriste votera l'amendement numéro un. Par contre si ce texte se résume essentiellement ce dispositif qui est de mon point de vue un amendement d'appel d'appel et et je reprends les arguments. De de notre collègue qui viennent de s'exprimer à un débat plus large à l'initiative du gouvernement et avec une participation active des collègues sénateurs pour la préparation du projet du de la prochaine loi de finances. Je crois que ça peut être un élément fort et un signal fort de maintenir une régionalisation d'une partie de la fiscalité sur les résidences secondaires comme ça a été proposé au départ dans ce texte, je crois qu'on ne pourra pas nouveauté la globalité du texte mais nous en voyons donc un signe d'ouverture de discussions forte sur ce sujet qui doit être associée à d'autres sujets liés à la fiscalité j'ai évoquais moi même dans mon intervention liminaire, le fait que il doit y avoir sur les multi-propriétaires de résidences secondaires, une fiscalité qui oblige une partie de ses propriétés à être mise sur le marché de l'allocation pour les résidences permanentes. Je crois que ce sujet-là doit être abordé en profondeur mais on envoie ainsi effectivement aux territoires en tension et à ce titre-là nous voterons donc majoritairement. L'amendement d'imbriquer tout en rejetant si effectivement la dimension régionale est confirmée. Parce que je ne crois pas que ce soit l'esprit que que nous défendons majoritairement ici au Sénat, qui défendons plutôt une dimension locales, départementales, régionales pardonnez départemental. Mais aussi à leurs collègues. Communal et intercommunal. Je vous remercie. Merci ma dernier. Merci monsieur le président je vais associé Denis Saint-Pé ma prise de parole. Je vais voter cet amendement j'avais voté le un amendement identique au PLF. Pour moi l'urgence de voter cet amendement, c'est de protéger les résidences primaires il y a des endroits où le mal est déjà fait, les, les taux de taxe d'habitation ont déjà augmenté pour les résidences secondaires et mécaniquement. La taxe foncière. Elle, elle a un effet sur les habitants. De au quotidien de de ces territoires et donc je veux ajouter aussi. Que pour 2023 la hausse des valeurs locatives va être telle que la taxe foncière va exploser et donc ça plus ça fait que pour les résidences primaires le va être insupportable. Donc il y a urgence à décoller. pour protéger les habitants des résidences privées. Primaire, les habitants de nos territoires. Merci. Merci cher collègue. Donc. Monsieur le rapporteur. monsieur le président. Mes, mes chers collègues. Effectivement, je partage l'intervention de ma collègue Christine Lavarde au revoir et réécrire donc là potentiellement la fiscalité locale à travers cet amendement. Alors je comprends la nécessité la frustration. L'urgence et c'est bien ce à quoi on va s'atteler dès les prochaines semaines. Je le je mais quand même, par exemple la corrélation ou la décorrélation c'est un des principes généraux du droit de la fiscalité locale. Faut-il l'évacuer tout de suite en cette matinée sans étude d'impact sans recul sans aller sur le terrain sans contrôle. Juste une petite question que je pose, même si j'en partage. J'en partage effectivement le le le doute. Voilà par ailleurs alors de d'une PPL sur les régions ont fini qu'un amendement sur le bloc communal et après on va parler des EPL. Est-ce que les régions sont en demande. Non, l'ARF a bien dit que non, il n'était pas je vous invite aussi à avoir une réflexion on reprendra à l'échelle de la PPL sur Lausanne quelle force voulons-nous donner collectivement sera dette qui va devenir de plus en plus le seul document qui va présider aux. Aux politiques publiques. En clair, les régions vont être chef de file de beaucoup de choses. Est ce que c'est ce que vous voulez, je vous invite à avoir du recul sur ce sujet en plus. Donc, on trouvera ça à travers Lausanne. Donc ce sera d'être contraignant ou pas et y compris en matière de politique publique du logement, en l'espèce, dès ce matin. À vous de voir. Est-ce que les EPL sont en demande cher Ronan Dantec j'ai réinterroger les EPL ce matin c'est pas aussi unanime que ça en fait, ce sont les APL les APL locaux du littoral qui sont très en demande ça c'est très juste mais pas les autres, les autres ils demandent effectivement à intervenir dans la mission de contrôle. Encore une fois qui va commencer dans les prochains jours et on aura l'occasion ensembles de d'évaluer réellement la demande en question est-ce que le bloc communal étant demande ce matin de décorrélation moi je ne sais pas ce qu'on les a interrogés, non. Est ce qu'on avait eu d'impact. Non je ne dis pas qu'ne sont pas des vrais sujets et des vraies questions. Je dis simplement qu'il faut prendre légèrement plus de temps. Alors les gens n'ont plus de temps, c'est pas le énième groupe de travail c'est quelques jours, quelques semaines pour le faire en réalité beaucoup plus sérieusement me croyez bien que je suis fort consciente donc rapporteur sur ce texte sur Lausanne de l'urgence à réinventer une fiscalité locale verte. J'en suis bien le 1er à le dire. Monsieur le rapporteur. Monsieur le président Gontard.

pas c'est pas un texte sur les régions sur la fiscalité, sur la fiscalité régionale et puis surtout de quoi on est en train de parler. On est en train de parler de l'amendement numéro un justement qui réécrit en partie qui écrit en partie le texte et qu'il le réécrit vraiment sur je dirais une urgence absolue. Alors quand vous dites que vous savez pas ce que peut penser le bloc communal de cette décorrélation il me semble qu'on est quand même les représentants des territoires et moi s'il y a quelqu'un ici qui m'explique que c'est pas une demande, une demande forte qu'on voit sur l'ensemble des territoires. Alors là j'y comprends plus rien et que ça soit dans les zones touristiques parce que effectivement c'est quelque chose qui est très prenant dans les eaux touristique mais pas que dans les zones touristiques. Moi je suis en Isère, oui sur les stations de ski, on a cette problématique qui est très forte mais pas que sur des zones rurales et très rurales de montagne, on a cette problématique pour arriver à vivre sur nos territoires pour pouvoir faire en sorte que des jeunes puissent accéder. À un logement à à des à des prix qui ne s'envole pas et donc évidemment que c'est une demande très fort de l'de l'ensemble des des élus cette décorrélation et puis derrière ça il y a aussi cette autonomie financière qu'on a enlevé et qu'on continue d'enlever à l'ensemble des collectivités et des communes sur notre territoire. Donc moi je ne comprendrais pas que ici. Notre assemblée ne votent pas cet amendement. Et du coup oui c'est une réécriture de texte et derrière votre ce texte parce qu'il y a une urgence, il y a un appel très fort qu'on doit faire auprès du auprès du gouvernement, rien que par ça, ça se justifie. Merci. Si cher collègue donc j'ai été saisi d'une demande ce scrutin public. Monsieur le Ministre. Étant. Un, un mot parce que c'est vrai que c'est un débat très intéressant que vous avez déjà eu. Lors du projet de loi de finances de 2023. Ça été rappelé. Vraiment on est très à l'écoute de cette problématique, réelle je voudrais rappeler malgré tout que le fait de supprimer la taxe d'habitation sur les résidences principales. Augmente de fait la différence de fiscalité entre les résidences principales et résidences secondaires et d'autre part la majoration sur les résidences secondaires de la taxe d'habitation est décorrélé de toute augmentation d'impôts locaux jusqu'à 60% je le rappelle, pardon, oui en zone tendue dans les zones dont on parle bien sûr dans les zones dont on pas. En zone tendue et d'autre part, on est tout à fait ouvert et c'est ce qui a été prévu dans le projet de loi de finances 2023, revoir la cartographie ce qu'est le travail qui est en cours qui est qui est conduire en concertation avec les associations d'élus et très rapidement le décret le plus rapidement possible. Le décret sera publié pour vous permettre permettent aux collectivités locales aux communes d'augmenter leurs taxes. Pour celles qui seraient concernés par la, la nouvelle carte avant le premier octobre 2023 pour une fiscalité 2024. Merci, monsieur le Ministre, le président Roquier.

sont 12 élus surtout du territoire donc qu'il y a des maisons ici et les mêmes. Les maisons secondaires, soit ne sont pas élus au conseil municipal. Alors la tentation pourrait être, je veux dire on monte pas

Et chers collègues donc j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur l'amendement numéro 1 à l'article 1er de la proposition de loi. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable. L'avis du Gouvernement est défavorable, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par article 56 du règlement de ce que tu

Le scrutin est clos. Le résultat du scrutin. Nombre de votants, 344. Nombre d'exprimer, 318 pour 153 contre 165, le Sénat n'a pas adopté. Alors je mets aux voix l'article 1er. Qui est pour l'article 2 Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Il y a un article additionnel après l'article 1er, l'amendement de Madame briquet. Merci monsieur le président. La part des deux ça déjà été dit la part des ménages propriétaires de leur résidence principale 58% ne progresse plus. Depuis 2010, alors que dans le même temps le nombre de résidences secondaires et de logements occasionnels augmente plus vite que l'ensemble du parc et cette hausse s'est accentuée sur les 5 dernières années en ne traitant pas ce sujet ont laissé s'installer un sentiment d'abandon d'injustice et une incompréhension profonde. Particulièrement chez les jeunes générations. L'amendement proposé par notre groupe répond à la problématique soulevée par la présente, proposition de loi, il vise à étendre la possibilité de majorer le plafond de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à toutes les communes qui le souhaitent, pas seulement en salle le situé en zone tendue. Cela permettra d'ouvrir cette possibilité dans des zones moins denses mais qui sont néanmoins. Par le Par le phénomène des résidences secondaires. C'est notamment le cas de certains territoires ruraux au détriment des populations vivant dans ces territoires, cela va aussi dans le sens du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales en leur laissant le choix de majorer ou non cette Dax, faisons confiance aux maires. Il propose également de permettre de majorer jusqu'à 100% au lieu de 60 pour ça. Actuellement, le plafond de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Cette recommandation a été faite par le Conseil des prélèvements obligatoires. Dans son rapport sur la fiscalité locale dans la perspective Dusan du 25 octobre 2002, Merci monsieur le rapporteur. À travers chaque projet de loi de de finance qui propose donc que la majoration puisse aller jusqu'à 100%, c'est-à-dire que la part communale de la taxe d'habitation, pourrait être. Doublé pour rappel c'est 60% aujourd'hui. Cette majoration de HRS. C'est une façon de. j'ai lu aussi le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires. a proposé d'élargir le périmètre de la tu élevés et de la majoration de la sécheresse, tout en les limitant aux zones tendues. Alors que cet amendement propose. De l'étendre aux zones rurales. La proposition de CPO était mise en, en oeuvre par ailleurs dans la loi. De finances. je permets de vous rappeler la position de la Commission exprimé la semaine dernière, qui est de voir d'abord comment s'applique l'extension du zonage proposé par la loi de finances, on l'a déjà dit, je le redis, sans procéder à des augmentations de fiscalité dans les faits est difficilement. Mesurable. Donc ce sera un avis de retrait sinon défavorable. Si Monsieur le Ministre. Même avis même avis. Donc je mais aux voit cet amendement. De avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre.

Merci Monsieur le Président, l'objet de cette du président roumain, demande de notre groupe et d'élargir le dispositif optionnel proposée à l'assemblée des territoires un hexagone et dans les outre-mer quand sa rédaction actuelle le limite à un nombre réduit de communes dont la liste n'est pas d'ailleurs à ce jour connu dans connu dans l'attente d'un décret d'application. La perspective d'ouvrir une possibilité de taxation au bénéfice des établissements publics Fangio est intéressante aux yeux des auteurs du préférant amendement il convient cependant d'en accroître la portée pour permettre une réelle effectivité de l'article. Telle est l'objet du présent amendement. Merci monsieur le rapporteur. difficultés importantes posées par l'article 2 qui elle est l'inégalité de traitement entre les contribuables puisque la taxation serait différente selon que le logement est situé dans un périmètre d'un EPF local ou d'État. Je m'attendais à ce qui les amendements pour corriger cet, cet aspect-là des choses entre PS local et et l'État. Mais ça n'est pas le cas. En outre, il crée une taxe en dans les zones non denses. Alors que la situation des résidences secondaires n'y avait pas du tout la même. Dans bien des endroits, les résidences secondaires sont plutôt vu comme des sources d'attractivité. Ça a été dit oui que c'est extrêmement complexe à appréhender mais on est tous, on sent de la nécessité d'un débat et d'agir et les moyens d'entretenir le Patrimoine bâti. Alors cette taxe serait décidé non par la commune, mais par un EPF qui pourrait donc aller à l'encontre des choix de politique du logement fait par la commune. Donc en cohérence avec la position de la Commission défavorables à l'ensemble de la proposition de loi, je ne peux qu'avoir un ami un avis. Défavorable. Merci Monsieur le Ministre. Même avis défavorable. Monsieur Dantec. Oui. Une des raisons pour lesquelles nous sommes restés sur les zones tendues, c'est aussi par rapport à ce principe de constitutionnalité. Même si on est alors vraiment plus dans le confiscatoire, perdu la région Véro qui a plus que 25%. Et toujours de manière optionnelle, je le rappelle. C'est pour ça qu'on est resté sur les zones tendues, où la question se pose. Totalement et où à mon avis en terme de constitutionnel, il n'y aura aucune difficulté puisque l'État reconnaît lui-même la difficulté sur les zones tendues, c'est pour ça qu'on en est resté aux entendu. Un 1er point 2ème point et là je m'étonne un peu des propos du rapporteur qui dit mais finalement les EPFL sont pas tous d'accord là-dessus dessus vous avez tous reçu un courrier du réseau des EPFL soutenance elle proposition les EPFL aujourd'hui sont très demandés par les communes, par les intercommunalités. C'est le cas en Loire-Atlantique, c'est le cas un peu partout et elles ne peuvent pas répondre à la demande qui est absolument centrale et qui va augmenter avec Lausanne. Donc là on est sur un consensus et je le rappelle et c'est pour ça qu'on en est resté aux établissements publics fonciers locaux que ce sont les élus locaux qui décident dans les établissements publics fonciers locaux rien, personne d'autre, donc c'est bien. Le bloc communal qui décide. Donc là on est vraiment dans l'autonomie fiscale des des communes. 2ème point dernier point en terme de recettes. Je crois que c'est moi qui a dit, mais à un moment il faut quand même des recettes. Oui, il faut des recettes. Soit les EPFL vont augmenter le taux. Pour la totalité des taxes, taxe d'habitation, taxe sur les résidences secondaires et contribution économique soit elles limitent leur augmentation parce qu'elles ont besoin de recettes aux résidences secondaires. C'est ça le choix qui est sur la table, soit elles vont augmenter, tout le monde. notamment la fiscalité économique soit elles augmentent uniquement en zone tendue ce qui participe de la déstabilisation du marché qui sont les résidences secondaires. C'est ça la logique de de de ce texte aujourd'hui effectivement c'est soutenu par les EPFL s'est décidé dans tous les cas que par le bloc communal et les élus locaux. Je ne vois pas de raison de pas de le vote le côté collectivement.

pas cette ce retour concernant tous les autres EPF et compris État régions qui ont une approche différente qui met et sans compter les zones blanches, il faudrait qu'on si on se penche véritablement le là dessus. Et puis concernant les le fonctionnement des EPF il fonctionne à partir de dotation de crédits budgétaires de l'État de dotation pour l'instant on n'a pas un État ou un retour concernant des baisses de ces dotations à la suite de la TSE, si vous voulez. Donc à ce stade là de l'histoire,

qui est de soutenir l'Intelligence des maires et des présidents d'Interco dans les décisions et donc de leur donner de l'autonomie et j'avoue que je suis parfois surpris que notre assemblée ne le fasse pas ma 2ème remarque c'est pour remercier le Monsieur le Ministre de ses explications détaillées sur les motifs de ces avis, c'est en effet toujours très intéressant parce qu'au fond, voilà notre rapporteur qui je le sais partage cette idée de donner plus de moyens, même s'ils souhaitent plutôt retardé les décisions pour les globaliser dans les examens Dusan et d'autres sujets et paradoxalement, il se trouve à défendre une position qui a été celle du gouvernement et à discuter d'un sujet les dotations des EPFL les EPFL nous disent qu'ils sont inquiets sur leur capacité à agir parce que centre-ville than. Résidences secondaires, exigence de construire nécessite des moyens dont ils ne disposent pas avec les dotations actuelles. Nous, nous ne disons pas on augmente la fiscalité, nous disons, nous donnons au maire, au président Interco aux élus qui siègent dans les EPFL la possibilité de bénef de choisir eux-, mêmes les politiques qu'ils entendent mener sur leur territoire. Et je pense que cette mesure mérite l'attention et même le soutien sur tous les bancs de cette assemblée.

Qui est contre. Qui s'abstient.-il être adopté. Donc je mais aux voix l'article 2. Qui est pour l'article 2. Un vote qui est contre. Qui s'abstient-il être adopté. Donc je vais mettre aux voix l'ensemble du texte qui ne comprend plus que l'article de puisque l'article 1er n'a pas été voter. J'ai été saisi d'un une demande de scrutin public. Par le groupe Les Républicains sur l'ensemble de la proposition de loi. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 de règlement. Le scrutin est ouvert.

Tous les orateurs l'ont dit. La situation est grave mais peut-être pas désespérée. Elle est. Et on doit trouver des solutions urgentes. Je voudrais sur l'examen de cette proposition de loi rappeler plusieurs éléments qui viennent appuyer les intentions de ce texte qui a le mérite de poser cette problématique. Si nous avons entendu les réticences au dispositif qu'il prévoit, j'aimerais que nous ayons collectivement conscience que nous nous pourrons sans cesse reporter un débat essentiel et nécessaire en septembre temps des mesures réelles visant à juguler les problèmes évoqués. Nous ne pouvons de manière répétée convenir unanimement au sein de cet hémicycle, que le problème est réel et pourtant ne pas agir. Les habitants de nos régions sont menacés et je crois que notre chambre aurait honneur à être à l'initiative d'un vrai débat porteur de mesures vertueuse pour nos territoires et leurs habitants. Le problème est d'autant plus large que les flux démographique s'accentue à destination des régions concernées augmentant entre autres les problématiques de logements pour les locaux. Défendre le droit de vivre au pays, c'est éviter l'exode irrémédiable et le déracinement des populations attachés à leur terre. Porteuse de leur culture et de leurs traditions. Cela serait préjudiciable à la richesse même de nos régions que nous aimons tant, a rappelé, si je prends le cas de la Corse elle conjugue depuis plusieurs années à la fois un des taux les plus forts de résidences secondaires, 40% en général 60% dans les zones touristiques, couplé à un afflux démographique important équivalant à un tiers de la population sur les 25 dernières années. Cette situation pèse lourdement sur le logement et engendre une spéculation effrénée à laquelle se greffe une insuffisance des infrastructures inadaptées à un tel afflux. Capacité d'accueil sanitaire sous tension, ressources en eau rediriger de l'agriculture vers les zones d'habitation dessalement de l'eau de mer saturation de la gestion des déchets. Voilà. En bref, l'ensemble des questions plus larges que ce débat pour donc leur faire que notre responsabilité politique nous engage à résoudre de manière consensuelle et vertueuse. Je vous remercie.

Le scrutin est clos. Alors. Les résultats du scrutin, le nombre de votants, 343. Le nombre d'exprimer, 326 pour 77 contre 249, le Sénat n'a pas adopté. Je vais suspendre la séance pour quelques instants afin de laisser au gouvernement, le temps de s'installer pour la suite de l'examen du texte. La séance est suspendue.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale visant à réhabiliter les militaires fusillés pour l'exemple. Durant la première guerre mondiale à la demande du groupe écologiste solidarité et territoires. Dans la discussion générale. La parole est à madame Patricia Mirallès, secrétaire d'État chargé des Anciens combattants et de la mémoire. Monsieur Monsieur le président, monsieur le président de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées. Monsieur le rapporteur. Mesdames les sénatrices messieurs le sénateur. Votre assemblée réunie pour examiner la proposer de la proposition de loi visant à réhabiliter les militaires fusillés pour l'exemple. Durant la première guerre mondiale. Dès la fin de la guerre. Les assemblées parlementaires de la République ont consacré un temps considérable à cette question, oh combien sensible et complexe. Elles ont fait. Dans des débats qui ont toujours transcendé les clivages politiques arrive s'il joue. Notre rapport à l'injustice. Et parce que cette question. Personne. Ne peut prétendre à avoir le monopole. De l'émotion. De quoi parlons-nous. En effet. De 639 militaires condamnés à mort par des conseils de guerre et fusillés et dans les archives en garder la trace. Dans leur très grande majorité ils furent exécutés dans les deux premières années de la guerre, condamné par la justice militaire d'un pays placé au bord du gouffre et qui dans une forme de panique. Face à des revers jugée inexplicable. Exiger dans le consensus social d'alors la sévérité. Il y a parmi eux. Des tiré au sort. Et cette exceptionnellement révoltant. Mais ce fut exceptionnellement rare aussi et ceux-là ont été réhabilité par la Cour de cassation ou la cas ou la cour spéciale de justice militaire. Ce n'est plus de dont nous débattons aujourd'hui. Que cette sévérité se soit traduite dans bien des cas par l'application d'une force injuste de la loi, nul ne peut le constater aujourd'hui. Les contemporains. Les frères d'armes des militaires exécutés comme parlementaire et parfois les 2 à la fois. S'en sont émus. Alors le travail des historiens ne le dit. Les plus hautes autorités de la République l'ont reconnu. C'est le 1er ministre Lionel Jospin en novembre 1998 à Khan au pied du Chemin des dames. Demandant. Que ces soldats, fusillés pour l'exemple au nom d'une discipline dont la rigueur n'avait d'égale que la dureté des combats. Réintègrent aujourd'hui pleinement notre mémoire collective nationale. C'est le président de la République Nicolas Sarkozy, 10 ans plus tard qui veut penser aussi. À ceux qui n'ont pas tenu à ceux qui n'ont pas résisté à la pression trop forte. Ah l'horreur trop grande et qui un jour a tant de courage tente d'héroïsme ce sont. Resté paralysé au moment de monter à l'assaut. Je penserai à ces hommes dont on avait trop exigé. Qu'on avait trop exposés que parfois des fautes de commandement avaient envoyé au massacre et qui un jour n'ont plus la force de se battre. 90 ans après la fin de la guerre. Je veux dire au nom de la nation que beaucoup de ceux qui furent exécutés alors ne s'étaient pas déshonorés n'avait pas été des lâches et plus simplement ils étaient allés jusqu'à jusqu'à l'extrême limite de leurs forces et il poursuit, je veux dire que la souffrance de leur épouse et de leur époux. Fut aussi émouvante. Que la souffrance de toutes les veuves et de tous les orphelins de cette guerre impitoyable. Souvenons-nous qu'ils étaient des hommes comme nous. Avec leurs forces et leurs faiblesses. Souvenons-nous qu'ils auraient pu être nos enfants. Souvenons-nous qu'ils furent aussi des victimes d'une fatalité. Qui dévore attendent d'hommes et qui n'étaient pas préparés à une telle épreuve. Mais qui aurait pu l'être. C'est le président de la République François Hollande à Cerny en aloi en 2017. 100 ans après, il ne s'agit plus de juger. Il s'agit de rassembler. Tous, c'était des soldats. Ils aimaient leur patrie. Il voulait la défendre comme les autres. Ils n'étaient que des hommes faillibles. Comme tous les hommes confrontés à la démesure d'une guerre sans limite leurs souvenirs appartient aujourd'hui à la nation. nation. Il existe aujourd'hui un large consensus historique sur les faits, le travail des historiens a permis de, de l'établir. À chacun peut accéder aux sources grâce à la décision du président Hollande de rendre disponible en ligne. Toutes les archives de ces procédures. En lisant les jugements parfois sommaires. Des conseils de guerre comme les archives des procès en révision et en réhabilitation on comprend. Que la part laissée à la défense avait été faible. Qu'il y avait fréquemment pas eu d'instruction, et que trop souvent les témoins n'avaient été ni recherché ni entendu il y a aussi un large consensus sur la mémoire. On a indubitablement juger des hommes dont la volonté avait été abattu par la violence des combats dans la violence, la volonté avait été aboli et qu'aujourd'hui le soigneur et car l'on connaît maintenant les syndromes post-traumatique, les effets des bombardements intensifs qui peuvent rendre fou. Qui paralyse. Oui. Il faut faire mémoire de ses hommes. Mais on ne peut le faire. Dans n'importe quelles conditions. Le législateur doit voir le passé mais aussi se projeter dans l'avenir. Il est celui qui donne à notre état de droit, ses contours. Alors pourquoi écarter cette proposition de loi en l'état. Pour maintenir un 3ème consensus celui sur la méthode. Les assemblées qui dans les années 20 et 30 ont débattu des jugements prononcés par les conseils de guerre et les moyens d'y revenir ont débattu des lois d'amnistie de de de révision n'ont pas dévié d'un principe. À une condamnation individuelles ne pouvait répondre qu'une réhabilitation individuelles pourquoi. Parce qu'elles ont voulu respecter le principe de séparation des pouvoirs. Et que leurs membres avaient conscience que certaines condamnations n'était pas contestable. Jean-Marc Todeschini qui connaît si bien le sujet et à qui la mémoire des fusillés doit tente depuis 1998. Rappelé devant l'Assemblée nationale en 2016. Une réhabilitation générale poserait problème. La plupart des fusillés pour l'exemple été condamnée par l'arbitraire, voire l'aveuglement d'une justice militaire expéditive. Cependant tous les procès n'était pas expéditive ou arbitraire, certaines condamné l'ont été hélas pour de bonnes raisons certaines accusations ne souffrait pas de contestation. Il ne faut pas que les revendications parfois légitimes des associations prennent le pas sur tout, et même sur la justice, ce serait consacrer une forme d'arbitraire. On ne peut répondre à une injustice par une autre injustice un arbitraire par un autre arbitraire, même quand on est persuadé que la justice et de son côté. Alors oui. Regardant l'histoire en face, mais ne cédons pas de tentation également dangereuse. La réécrire ou rejugé. Il nous faut à la fois reconnaître. Que beaucoup de ces fusillés mérite d'être réintégré dans notre mémoire nationale. Mais que ce principe de reconnaissance poser la diversité des situations individuelles appartient aux historiens pas au législateur. Et qu'en plus d'un siècle de distance, elle appartient pas davantage au juge. Or dans le texte adopté par l'Assemblée nationale on ne t'en as rejugé par le mec mais le mécanisme d'abord de la réhabilitation générale collective civique et morale. La réhabilitation. Elle a, elle est du ressort de la justice. Passée cette limite. N'est-ce pas empiéter sur le principe essentiel de l'organisation de la République auquel il est inconcevable de déroger. La séparation des pouvoirs par l'inscription sur les monuments aux morts ensuite car cette entrée dans le chat d'implication de l'article L. 515 tirer un du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre c'est de facto accordée à tous ces condamné la reconnaissance qu'ils sont morts pour la France. Mais nous butons de nouveau sur le fait que tous n'étaient pas innocent. Ces 2 dispositions heurte donc notre droit comme elle heurte une partie importante des associations d'anciens combattants. Peut-on vraiment réussir à apaiser les cicatrices du passé en braquant une large partie du monde combattant qui nous observe aujourd'hui. La proposition de loi laisse aussi des zones d'ombres sur la procédure et cela rejaillira sur les mers. Qui leur dira si le fusiller dans les descendants ou une association demande d'inscription du nom sur le monument de leur commune. Était bien l'un des 639 dans la demande de révision n'a pas été rejeté dans les années 20 ou 30. Les maires devront-ils faire leurs recherches. L'administration ou la justice devront-t-elle répondre à leurs interrogations. La proposition de loi ne le dis pas. cadre d'une procédure d'une procédure qui est collective. Face à l'hétérogénéité des cas individuels. Un doute ne pèsera-t-il pas sur le rétablissement de leur honneur. Cela vous laisse de voix. Rejeté la proposition de loi. Non pas pour rejeter la la mémoire des fusillés dans l'innocence n'a pu être établi mais pour rejeter les effets généraux et problématique de ce texte ou amender car je tiens. À vous mettre en garde contre l'adoption de ce texte en l'état. Ne prenait pas le risque de son adoption, sous le coup d'une légitime émotion. Vous pouvez en retirer ce qui divise est entré de plain-pied dans la réintégration mémorielles pour donner aux paroles qui se succèdent depuis 25 ans. La force de la loi. C'est ce que fait l'amendement déposé par André Gattolin du groupe RDPI et je tiens ici à saluer de manière appuyée le travail que le président Patriat et lui ont conduit dans la recherche d'une voie de compromis dont je sais qu'elle satisfait le monde combattant et qui vous offre l'opportunité d'adopter un texte de conciliation. Et de réconciliation. Je vous remercie. Merci madame la ministre. Mes chers collègues, je vais sur. Pour la séance elle sera reprise à 14h 30 pour la suite de l'examen de ce texte. La séance est suspendue.